Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Jean Louis Debré. Évoquer Jean Louis Debré, c’est honorer la mémoire d’un grand serviteur de la V République. Son père, Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, père de la Constitution, lui transmit les valeurs du gaullisme, auxquelles il restera attaché toute sa vie sa vie et qu’il défendra aux côtés de Jacques Chirac. Élu député de l’Eure en 1986, il siégea en même temps que son père et son frère à l’Assemblée nationale. Ce fut pour cet amoureux de la République une grande fierté. Il fut aussi maire d’Évreux. Ministre de l’intérieur de 1995 à 1997, il dut faire face aux attentats terroristes que subit alors notre pays. Président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007, il s’attacha à renforcer la fonction de contrôle du Parlement, mais aussi le respect du statut de l’opposition. Le fils de celui qui fut le père de la Constitution veillera à ce qu’elle soit appliquée avec la plus grande rigueur. Présidant le Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, Jean Louis Debré s’est attaché à ce que puisse être adoptée et que se déploie la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.

Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille et à ses proches. Mes chers collègues, le 27 février dernier, nous avons appris, avec colère et tristesse, le décès de notre compatriote Ohad Yahalomi, enlevé, puis retenu à Gaza depuis le massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Comme de trop nombreux otages, il ne reviendra pas auprès des siens. Nous pensons à ses proches, à son épouse et à ses enfants particulièrement. Nous avions, cher Roger Karoutchi, rencontré sa famille à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour lui dire notre soutien.

qui nous fait l’honneur d’être présent pour cette séance consacrée à la situation en Ukraine et à la sécurité en Europe. J’ai le plaisir de saluer également en tribune d’honneur le président du Parlement d’Estonie, M. Lauri Hussar, accompagné d’une délégation de quatre parlementaires. Nos collègues Édouard Courtial, président du groupe d’amitié France Pays Baltes, et Rémi Cardon, président délégué Nous avons pu aborder, avec nos homologues du Parlement estonien, des sujets aussi essentiels que l’avenir de la relation transatlantique, les défis énergétiques et de sécurité auxquels nos pays sont confrontés, particulièrement l’Estonie, lors de l’audience à laquelle à laquelle ils ont pris part avec nos collègues Loïc Hervé, vice président chargé de la coopération interparlementaire et des groupes d’amitié, Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et Jean François Rapin, président de la commission des affaires européennes.

Face aux menaces sur l’avenir de la sécurité collective en Europe, la sécurité de l’espace baltique constitue un enjeu d’une importance cruciale. La France et l’Estonie, dont les relations diplomatiques sont plus que centenaires, y contribuent activement par leur étroite coopération dans de nombreux domaines, dont celui de la défense, dans le cadre européen comme dans celui de l’Otan. Je pense particulièrement, en cet instant, à nos aviateurs et soldats qui sont présents sur la base de Tapa. La diplomatie parlementaire – en particulier celle du Sénat – joue également un rôle actif dans les excellentes relations qu’entretiennent nos deux pays. permettez moi de souhaiter à nos amis membres du Parlement estonien la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française, mais aussi de leur

M. Philippe Bas ayant été nommé au Conseil constitutionnel, son mandat de sénateur a pris fin le 1 mars 2025 à minuit. Par lettre en date du 28 février 2025, le ministère de l’intérieur m’a fait connaître que, en application de l’article L.O. 320 du code électoral, M. Bas était remplacé par M. David Margueritte,

Le premier mot qui vient à l’esprit, lorsqu’on pense à lui, est celui de républicain. Il avait des formules assez drôles. Ainsi, lui qui était le fils de Michel Debré disait régulièrement qu’il était le frère de la Constitution de la V République, puisque Michel Debré était le père ci. Évidemment, la proximité entre cette œuvre majeure et la personnalité de Michel Debré était profondément marquante.

Il portait sur le monde, et notamment sur le monde politique, un regard amusé, ironique, informé. Il n’était guère de secret qu’il ne connût, mais cela n’empêchait pas l’indulgence qu’il avait non seulement envers ses collègues engagés en politique, mais aussi à l’égard, au fond, de la nature humaine.

De son passé de juge d’instruction, il avait retenu bien des intrigues et bien des tics de personnalité, dont il faisait la matière de ses romans policiers. était un homme attachant et respecté. À la présidence de l’Assemblée nationale comme à celle du Conseil constitutionnel, il a fait la preuve de ses qualités humaines et politiques.

à ses enfants et petits enfants. Il était un homme que nous regrettons déjà.

situation, vous le savez, évolue d’heure en heure et nous place devant des responsabilités et face à des rendez vous que nous ne pouvons pas éluder. Hier encore, nous en étions au choc qu’a constitué, pour beaucoup d’entre nous, l’épisode du rendez vous, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche,

avec nous beaucoup de Français – et même une majorité d’entre eux –, nous avons ressenti la manière brutale et méprisante avec laquelle le président des États Unis a traité le président de l’Ukraine comme une offense à une certaine idée que nous nous faisons du respect entre États, entre responsables d’État, mais aussi du respect de principes et de valeurs auxquels nous sommes profondément attachés et auxquels nous pensions que les États Unis, notre allié depuis la Seconde Guerre mondiale, étaient aussi profondément attachés que nous le sommes.

des centaines de milliers de blessés, et – on a peine à l’évoquer dans un discours officiel – 20 000 enfants qui ont été déplacés pour que soit changée, par l’influence, leur identité ukrainienne, pour qu’elle soit abandonnée. Cette déportation est, pour nous, un crime contre l’humanité. Enfin, des centaines de milliers d’Ukrainiens, de femmes et d’hommes, ont été déracinés. Au fond, ils sont le visage de tout un peuple qui souffre. L’Ukraine souffre pour une raison extrêmement précise et datée : le 24 février 2022,

et pour écarter les responsables publics que le peuple ukrainien s’est choisis, et qui font preuve d’un héroïsme tout à fait remarquable.

À cet instant, il a été le visage de l’Ukraine, le défenseur de l’honneur de la démocratie, et il portait en même temps une partie de notre honneur européen. Le président Zelensky a honoré la mission qui est la sienne. Nous nous sommes sentis profondément solidaires de son refus de se plier à ces injonctions. Il y avait Il y avait eu bien des signes avant coureurs avant coureurs avant ce rendez vous de vérité et de dévoilement des intentions du président américain. Il y avait eu, d’abord, bien des rodomontades : l’annonce selon laquelle il pourrait régler le conflit ukrainien en un jour, par un claquement de doigts. Il y avait eu des déclarations extraordinairement inquiétantes au regard du droit des nations, avec l’affirmation selon annexer le canal de Panama, que les États Unis pourraient se rendre maîtres du Groenland, que, pourquoi pas, le Canada devrait être, à son tour, intégré aux États Unis et enfin que Gaza pourrait être placée sous contrôle de l’administration américaine.

que les rodomontades se transforment en actes. Et nous avons vu, très vite, un changement incroyablement inquiétant et extrêmement profond de la diplomatie américaine, puisque la semaine dernière, aux Nations unies, les États Unis ont voté avec la Russie et la Corée du Nord pour repousser une résolution dans laquelle était mentionnée la responsabilité de la Fédération de Russie dans la tentative d’annexion de l’Ukraine. Que les États Unis refusent de nommer l’agression dont l’Ukraine est victime a été, pour beaucoup d’entre nous, une prise de conscience. Il y a eu ensuite l’agression dans le Bureau ovale et les mots que le président Trump a utilisés. Je vous rappelle la phrase la plus significative : « Trouvez un accord avec Poutine ; autrement, nous vous laisserons tomber. indépendante, souveraine, soumise à la pire des menaces, une menace sur son existence même, et qui est abandonnée par le pays qui fut le leader de l’alliance des libertés cela est, pour beaucoup d’entre nous, extrêmement violent. Au fond, la question se résume assez simplement : si la Russie arrête les combats, c’est la guerre qui s’arrête si l’Ukraine arrête les combats, c’est l’Ukraine qui disparaît. Cette réalité si lourde et si choquante, il est très important qu’elle soit rappelée aujourd’hui, devant le Sénat de la République. a été annoncée une décision que beaucoup redoutaient, mais dont chacun voit les implications : l’annonce selon laquelle les États Unis stoppaient désormais les livraisons d’aide à l’Ukraine. Car le mot « suspension » ne trompe personne la suspension, dans la guerre, de l’aide à un pays agressé, cela signifie qu’on abandonne celui ci et qu’on accepte – ou qu’on souhaite – que son agresseur l’emporte. agresseur l’emporte. Pour la France, pour nous tous, pour les Européens et pour tous ceux qui sont attachés aux libertés et aux droits, pour ceux qui sont attachés à la Charte des Nations unies, par exemple, c’est évidemment tout à fait insupportable. Que ce soit un pays membre du Conseil de sécurité des Nations unies, c’est à dire garant de l’ordre international que les Nations unies incarnent,

guerre. Cette alliance que nous avons construite autour des États Unis reposait, comme énoncé dans la Charte, sur la primauté du droit du droit sur la violence. Je cite presque exactement la Charte des Nations unies : c’était le refus de la violence pour régler les conflits, c’était le droit du plus juste contre le droit du plus fort. C’est ce monde là que nous avons abandonné pour entrer dans un autre monde où, au fond, les principes sont abandonnés. Et cet abandon des principes menace l’existence même des relations internationales telles que nous les avons voulues et construites. C’est vrai de la guerre en Ukraine, mais c’est aussi vrai des relations commerciales et économiques, de l’idée que nous nous faisons du multilatéralisme, du fait que les grands ensembles du monde, à un égal degré de responsabilité, participaient ensemble à la définition d’un ordre mondial respectueux de ce que nous avons voulu et construit ensemble. Devant cette incroyable agression, cet abandon des principes et ce changement de l’ordre du monde, beaucoup d’entre nous, beaucoup de nos concitoyens, se trouvent désespérés. le message et la vision du Gouvernement, c’est que nous ne pouvons pas désespérer ! D’abord parce que nous sommes la France et que nous sommes l’Europe. Nous sommes l’Europe : cela signifie que, contrairement à ce que nous croyons ou à ce que nous laissons croire, nous sommes non pas faibles, mais forts, si nous comparons les capacités de l’Union européenne et les capacités de la Russie,

et nous ne savons pas qu’elle existe. Nos concitoyens pensent que nous sommes désarmés, mais je crois le contraire. J’ai en mémoire

» Ce que le général de Gaulle avait comme vision pour son peuple, ce peuple dont il avait la charge, nous devons l’avoir aussi pour l’Union européenne. Nous avons une force que nous ignorons

La responsabilité de l’Union européenne et des pays amis de l’Ukraine, c’est d’être capables de se substituer le plus rapidement et le plus efficacement possible aux livraisons américaines, de manière que l’Ukraine ne soit pas contrainte de craquer.

–, mais aussi tous ceux qui peuvent apporter leur aide à un pays qui se trouve devant une si grave menace militaire.

Il nous appartient de dire et de savoir si nous voulons être fidèles à cette tradition française. Cela entraîne plusieurs conséquences. La première d’entre elles est industrielle

les capacités de transport, la projection dans l’espace et le renseignement, nous sommes devant des responsabilités qui, de toute évidence, vont transformer notre manière d’être.

Des instruments de prêts sont préparés et un appel à l’épargne a été lancé, notamment en direction de la Banque européenne d’investissement (BEI).

La France a sans cesse déployé le drapeau de cet idéal dans les rangs de l’Union européenne. L’expression de cet idéal et de cette volonté politique est étroitement liée à la santé et au rayonnement de notre pays.

retrouver la capacité créatrice de notre pays et la confiance que nous devons avoir en nous mêmes – sont directement liées à la capacité d’influence que la France peut avoir sur l’Europe en portant un projet

Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce débat était indispensable, tant la situation est grave et lourde de conséquences pour notre pays. En quelques jours, l’Histoire s’est accélérée et les Européens sont aujourd’hui contraints de réagir dans l’urgence à la recomposition du paysage géopolitique. Le monde qui apparaît aujourd’hui en pleine lumière n’est pas nouveau dans son esprit ; c’est celui dans lequel l’humanité a baigné pendant l’essentiel de son parcours, celui où la force prime le droit et où les États ne peuvent compter que sur eux mêmes pour assurer la défense de leurs intérêts. Le Gouvernement a souhaité un débat sur la situation en Ukraine et la sécurité en Europe. Le sujet fondamental qui donne à la séance d’aujourd’hui toute sa gravité et son urgence est surtout la sécurité en Europe. La situation en Ukraine est bien connue. Ce malheureux pays, agressé par son voisin quatre fois plus peuplé, mène de façon héroïque un combat forcément inégal. Je veux dire ici de nouveau à M. l’ambassadeur d’Ukraine notre admiration pour le peuple ukrainien et notre respect pour les immenses sacrifices qu’il a consentis et qu’il consent encore, jour après jour, non seulement sur le front, mais aussi au cœur de ses villes, sous les bombardements quotidiens de l’agresseur russe.

vingts ans : la sécurité de l’Europe reposait avant tout sur la puissance militaire d’un pays non européen, les États Unis d’Amérique. Cette situation, due au contexte particulier de la guerre froide, s’est poursuivie trente ans après l’effondrement de l’URSS, dans l’illusion de ce que l’on a appelé « les dividendes de la paix ». Pendant trente ans, tous les pays européens se sont désarmés comme jamais ils ne l’avaient fait depuis qu’existent les États nations. Ce désarmement a porté, bien sûr, sur le format des armées, qui a fondu dans des proportions à peine croyables. Quelques chiffres : l’armée de terre est passée de 1 500 chars à la fin de la guerre froide à moins de 200 aujourd’hui, et de 400 pièces d’artillerie à 72. La saignée a été comparable, voire pire, chez nos alliés européens l’Allemagne est ainsi passée de plus de 4 000 chars en 1992 à environ 300 aujourd’hui, et de 3 000 pièces d’artillerie à une centaine au début de cette décennie.

Il faudra s’en souvenir avant de ressortir les rengaines pacifistes sur l’immoralité de toute exportation d’armement. La présidente de la Commission européenne a appelé dimanche à un réarmement rapide de l’Europe. Il faut saluer cette conversion récente des plus hautes autorités européennes aux vertus de la production d’armement, digne de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. On peut se demander si elle aura gardé le souvenir des débats qui avaient lieu encore récemment à Bruxelles sur la taxonomie : certains espéraient tout simplement interdire progressivement la vente, donc la fabrication des matériels de guerre, d’autres encourageaient les banques à ne pas financer l’industrie de défense. Très bien ! C’est l’élu du département le plus industrialisé de France qui vous le dit : ne sous estimons pas la gravité de notre affaiblissement industriel en matière de production de matériel de guerre, entre autres. Les compétences et les moyens de production qui ont été abandonnés ne pourront être restaurés d’un coup de baguette magique. Et puis, derrière les effets délétères des dividendes de la paix, il y a les effets psychologiques de l’effacement dans les consciences européennes de cet horizon des peuples que constitue la guerre, menace éternelle qui pousse les nations à se préparer, à se protéger, à anticiper et à se rassembler sur un socle de valeurs communes. La guerre était loin, elle ne concernait pas la vie quotidienne ; les questions de défense et le sens des priorités ont disparu du débat public. Tout cela explique la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, alors que la Russie accroît sa pression et que les États Unis ont annoncé réduire leur soutien et, surtout, le conditionner à une forme de vassalisation de l’Europe. L’alignement sur le narratif russe et l’espoir de faire de fructueuses affaires avec la Russie sur le dos des Européens sont, certes, des nouveautés de l’actuel président américain. Cependant, la dénonciation de la répartition inéquitable de l’effort de défense au sein de l’Otan et le pivot stratégique vers le Pacifique sont des constantes des administrations successives depuis la présidence d’Obama en 2011. Reste que nous, Français, avons toujours envisagé ce type de scénario. C’est ce qui a motivé notre choix de nous doter d’une capacité souveraine de dissuasion nucléaire. Les responsables français de l’après guerre, en particulier le général de Gaulle, ne voulaient plus jamais dépendre d’autres pays pour assurer la défense des intérêts vitaux de la France. Mes chers collègues, nous sommes désormais à l’heure des choix. Notre groupe politique considère que c’est ce chemin d’autonomie tracé depuis l’après guerre qu’il nous faut suivre à l’heure des périls. Cela suppose pragmatisme et ambition. Pragmatisme, car, avant de jeter le bébé américain avec l’eau saumâtre du bain trumpiste, il faut déterminer ce que les Européens peuvent encore raisonnablement espérer faire avec les Américains. Le Premier ministre britannique a indiqué, dimanche dernier, qu’un déploiement en Ukraine d’une force de maintien de la paix européenne après la fin des combats ne pourrait se faire qu’avec l’appui américain dans trois domaines : la logistique, les communications et le soutien aérien. Or rien de tout cela n’est acquis. Ambition, ensuite, car nous ne pouvons confier à d’autres pays notre destin. Je n’ai pas caché l’ampleur de la tâche, mais je ne veux pas non plus éluder nos nombreux atouts. La brutalité et les provocations du président Trump entraînent un véritable réveil européen, encore inimaginable il y a seulement quelques semaines. En témoignent les déclarations fortes du futur chancelier allemand, celles du Premier ministre polonais et celles de Kaja Kallas. Par ailleurs, l’Europe a les éléments de la puissance si elle est prête à les assumer : sa population, comme vous venez de le rappeler, monsieur le Premier ministre, et sa richesse économique, mais aussi certains points forts technologiques et scientifiques. En Europe, la France est écoutée sur ces sujets, car personne ne lui conteste la qualité et les capacités de ses forces armées. En outre, elle est le seul État doté de l’arme nucléaire au sein de l’Union européenne et le seul pays en Europe qui ne dépend en rien des États Unis pour la mise en œuvre de sa dissuasion. Sur ce sujet, il n’y a pas lieu de gloser sur l’épouvantail agité par les deux extrêmes quant aux prétendus risques de perte de souveraineté si le parapluie nucléaire français devait être étendu au territoire de l’Union européenne. Tout cela n’est guère sérieux, la dissuasion ne pouvant se partager. la question de savoir dans quelle mesure les intérêts vitaux de la France englobent certains éléments de la sécurité de l’Europe a depuis longtemps été évoquée par les présidents de la République successifs, le général de Gaulle en tête. Il n’y a pas lieu d’avoir sur ce sujet des débats oiseux, très éloignés de la réalité de la dissuasion nucléaire. Quant au rôle essentiel que la France doit jouer, il se justifie par notre promotion de l’autonomie stratégique européenne, par l’expérience, le professionnalisme et les capacités de nos forces armées, ainsi que par l’excellence technologique de notre BITD. Faisons prospérer ces atouts dans des partenariats concrets avec nos alliés européens. Naturellement, ces atouts auront peu d’importance si la France et l’Europe ne se lancent pas immédiatement dans un redressement historique de leur effort de défense. Nous avons le devoir de présenter aux Français la réalité telle qu’elle est, dans toute sa gravité et dans toute sa dureté. Mes chers collègues, nous sommes tous des élus de terrain. Comme vous, j’entends les préoccupations quotidiennes de nos compatriotes qui tournent autour du chômage, de l’insécurité, du recul et de la dégradation des services publics dans nos territoires. Pourtant, si nous devons redresser notre effort de défense, il faudra bien prendre l’argent quelque part n’éludons pas cette question très difficile ! L’État est financièrement exsangue. La solution ne peut venir d’un nouvel alourdissement de la dette, qui atteint des niveaux insupportables.

Je pense que c’est peut être là le point le plus important de notre débat : pourquoi la guerre en Ukraine concernerait elle chaque Français ? pourquoi devrions nous réarmer la France et l’Europe ?

Poutine poursuivra son projet, et nous connaissons déjà ses prochaines cibles : la Moldavie, la Roumanie, les États baltes, la Pologne et les Balkans occidentaux. Et c’est sans compter sur l’explosion de la guerre hybride que la Russie a déjà

Deuxièmement, si la Russie gagne la guerre en Ukraine, l’Europe enverra au monde entier un extraordinaire signal de faiblesse. Quel traitement espérer des autres puissances dans ces conditions ? Croit on qu’une Europe divisée, affaiblie et humiliée serait en situation de calmer l’appétit économique de Trump et des grandes puissances ? Oui, il va falloir accepter que la défense soit prioritaire par rapport aux autres politiques publiques, car si nous ne renversons pas le cours des choses, nous serons soumis et vassalisés. Dans ministre, il n’y aura plus lieu de parler de l’indexation des retraites, de la valeur du point d’indice ou de transition écologique, car la richesse nationale sera captée par d’autres.

Poutine ne respecte que la force. La seule chose qui puisse l’empêcher de commettre le pas de trop qui conduirait à un affrontement direct entre la Russie et les pays d’Europe, c’est l’aptitude des pays européens à être suffisamment dissuasifs. Nos capacités militaires sont donc notre propre garantie de sécurité. En conclusion, l’ensemble de la classe politique française va devoir faire face à ses responsabilités. Au risque d’être taxé de partialité, je crois que le Sénat peut montrer la voie dans ce domaine. Dans cet hémicycle, les divergences politiques et les désaccords, parfois profonds sur certains points, n’ont jamais empêché l’écoute de chacun et le respect mutuel. Je le rappelle, la loi de programmation militaire (LPM) de 2018 a été votée au Sénat par 96

C’est de ce consensus républicain que nous avons besoin dans ces heures graves. Je forme le vœu que tous les sénateurs puissent se faire l’écho dans leurs territoires de nos débats aujourd’hui, dans cet esprit de responsabilité et de gravité. Monsieur le Premier ministre, dans ce moment difficile, le Président de la République et le Gouvernement ne sont pas restés inactifs ; nous vous en donnons acte. Portons maintenant nos regards au delà, pour doter la France des moyens de défendre ses intérêts et la sécurité des Français, qui sont menacés, et diffuser en Europe notre volonté d’indépendance et de souveraineté. Oublions les vieux schémas de pensée, inadaptés à la situation grave dans laquelle nous sommes, et ayons le courage et la lucidité de regarder la dure réalité en face pour agir sans plus attendre : le temps nous est compté. C’est le sens de la conclusion que le général Beaufre tirait du drame de 1940 : « Les nations ne sont que les jouets du destin si elles n’ont pas su prévoir la montée des périls ni intervenir à temps pour les conjurer.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, « la guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées Les propos de Victor Hugo sont criants d’actualité : la véritable bataille se joue dans l’arène des convictions, des valeurs et des visions du monde. La guerre en Ukraine, au delà des affrontements physiques, est également une bataille des idées, où la démocratie, la liberté et la souveraineté sont en jeu face aux forces autoritaires et impérialistes. En effet, la guerre en Ukraine ne se limite pas à un simple affrontement militaire elle incarne un bras de fer idéologique et géopolitique pour l’avenir de la paix, de la liberté et de la démocratie. C’est non pas seulement l’Ukraine qui est en jeu, mais l’équilibre d’un monde en perte de repères. Alors que les menaces se font de plus en plus pressantes, résonnent en moi les premiers mots de l’hymne ukrainien La gloire et la liberté de l’Ukraine ne sont pas mortes. » Il nous faut prendre la mesure de ce qui se dresse devant nous. L’équilibre fragile que nous avons patiemment construit peut être anéanti, et tout ce qui a été édifié pour garantir la paix peut être balayé, car le retour de la guerre sur le sol ukrainien n’est que le prélude à une escalade qui semble désormais inéluctable. Nous ne sommes pas en guerre au sens traditionnel du terme, mais la guerre hybride a déjà commencé depuis plusieurs années ; c’est une réalité incontournable. Depuis plus de trois ans, le peuple ukrainien, avec une résilience inouïe, porte le poids de la guerre, affrontant des attaques militaires incessantes et une pression idéologique impitoyable. Il se bat non pas seulement pour sa propre survie, mais aussi pour des valeurs qui nous sont communes. Sa lutte est notre lutte. Nous devons affirmer notre solidarité avec ce peuple héroïque qui résiste avec courage. Combien de fois avons nous proclamé que l’Ukraine se battait pour nous, alors que nous devons nous battre avec elle ! L’Europe ne peut pas permettre que l’Ukraine soit sacrifiée dans des compromissions internationales qui l’excluent de son propre destin. L’Europe ne peut cautionner une sortie de crise qui priverait l’Ukraine de toute perspective, en entravant en premier lieu l’exploitation de ses ressources stratégiques. Nous ne pouvons pas tolérer qu’elle soit soumise à une domination à caractère néocolonialiste. Tout compromis privant l’Ukraine de son intégrité territoriale ou de son avenir européen serait une trahison pour l’ensemble de l’Europe.

Le vent de l’autoritarisme souffle fort aujourd’hui. Bien qu’antagonistes, ces puissances partagent des caractéristiques et des objectifs inquiétants étendre leur domination en divisant pour mieux régner, affaiblir notre démocratie, réécrire l’Histoire à leur convenance et étouffer la vérité sous le poids de la désinformation organisée.

dont nous devons tirer toutes les conséquences. Il nous faut nous ériger en défenseurs de relations internationales fondées sur la coopération, en défenseurs des organismes et des institutions internationaux.

Et pour Donald Trump, l’Europe n’a jamais été une alliée ; au mieux, une protégée. Trump voit le monde comme un immense jeu de Monopoly, avec ses transactions immobilières. Le traquenard médiatique du Bureau ovale a dévoilé la seule motivation de Donald Trump, que l’on peut résumer cyniquement ainsi : Cette nuit, il Cette nuit, il est allé encore plus loin en gelant l’aide apportée à l’Ukraine pour pousser à sa capitulation. Un sursaut est urgent. Seule une volonté collective, unie, pourra garantir à nos citoyens une paix durable et une Europe forte, prête à défendre ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Face à ce contexte mondial tumultueux, nous ne pouvons plus être des spectateurs passifs.

Les différends qui ont marqué la récente conférence de Munich sur la sécurité et la réunion convoquée à la hâte par Emmanuel Macron le 17 février dernier ne doivent plus avoir cours. Nous ne pouvons plus laisser les puissances russe et américaine semer la discorde parmi nous. L’autonomie stratégique européenne, loin d’être une chimère, doit devenir un objectif prioritaire. Il s’agit non pas seulement de renforcer nos capacités militaires, mais aussi de garantir notre indépendance numérique, économique et commerciale. Il est inconcevable que l’Europe demeure sous la tutelle des États Unis ou que des régimes autoritaires comme la Russie puissent exercer une emprise sur nos infrastructures critiques et nos informations. Seule une Europe ferme et déterminée, prenant son destin en main, pourra préserver sa souveraineté. L’inaction et l’absence de coordination servent avant tout les intérêts de Poutine et de Trump, qui, comme l’a justement

faut rappeler que l’Union européenne fournit un soutien financier globalement plus important que les États Unis, bien que ces derniers conservent un rôle de chef de file en tant que principal fournisseur d’aide militaire directe, influençant d’ailleurs ainsi fortement la stratégie militaire dans le conflit ukrainien. Ce dilemme budgétaire se noue dans un contexte où l’Europe fait face à de nombreuses autres menaces : cyberattaques, guerres hybrides invisibles, déstabilisation dans des régions stratégiques comme l’Arctique, du fait de ses ressources et de ses voies commerciales vitales. L’Europe se trouve à un carrefour crucial : doit elle continuer à financer l’Otan selon les exigences américaines ou bien investir davantage dans sa propre défense et sa souveraineté pour peser davantage au sein de l’Otan ?

Actuellement, près de 80 % de nos équipements militaires ne proviennent pas de l’Union européenne. Nous devons donc adopter une vision d’ensemble et œuvrer à ce que la reconstruction industrielle militaire aille de pair avec le renforcement de nos capacités d’intervention. À cet égard, la France porte une responsabilité particulière. En tant que puissance nucléaire et État membre clé de l’Union européenne, il lui revient de jouer un rôle central. En meneur audacieux, elle doit être le moteur de cette transformation européenne et défendre l’unité de l’Europe face aux défis géopolitiques actuels.

? de la position de la France et de sa participation au plan de 800 milliards d’euros pour réarmer l’Europe qui vient d’être annoncé aujourd’hui par Mme Ursula von der Leyen ? Français un discours de vérité. Annoncez clairement les sacrifices qui devront être faits pour résister aux nouveaux impérialistes. Annoncez clairement les conséquences qu’aura la guerre commerciale engagée contre nous par les États Unis. Nous devons – vous devez – repenser votre ligne politique à l’aune de cette nouvelle donne internationale. Notre contrat social ne peut pas être sacrifié sur l’autel de l’agression russe en Ukraine. D’autres sources de financement doivent être imaginées dans le cadre du patriotisme fiscal que vous devez affirmer, y compris envers ceux qui étaient présents le 20 janvier dernier lors de l’intronisation de M. Trump, Nous vous rappelons aussi notre proposition pour garantir notre sécurité nationale, défendre nos intérêts vitaux et répondre aux différentes difficultés de financement des entreprises du secteur de la défense. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a proposé la création d’un livret d’épargne dédié à la défense et à la souveraineté. Allez vous étudier cette solution ? par ailleurs la confiscation des 250 milliards d’euros d’avoirs russes pour financer la protection de l’Ukraine et de l’Europe ? Sur le plan diplomatique, en lien avec le plan financier que je viens d’évoquer, comptez vous revenir sur les mesures qui, depuis 2017, ont considérablement affaibli notre appareil diplomatique dans le monde ?

Sur le plan humain, dans le cadre d’un éventuel accord de paix pour l’Ukraine, sachant qu’il est impossible d’exclure toute reprise des hostilités, envisagez vous le déploiement d’une force de maintien de la paix sur la ligne de front du côté ukrainien dès l’arrêt des combats ? ? Enfin, sur le plan des sanctions, où en est la création d’un tribunal spécial chargé de poursuivre le crime d’agression commis contre l’Ukraine, soutenu par une coalition de trente huit pays, dont l’immense majorité des pays de l’Union européenne ? La guerre en Ukraine restera La guerre en Ukraine restera inscrite dans l’Histoire comme le témoignage incontestable de la défense d’une certaine idée du principe de souveraineté. Cet affrontement militaire doit se solder par le triomphe de la justice du droit contre la brutalité de la force.

Beaucoup ont éprouvé ce même sentiment de sidération vendredi, en voyant en direct le président Trump reprendre les éléments de langage de M. Poutine pour humilier le président Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Ces propos insultants contre la politique internationale des États Unis d’Amérique menée par les prédécesseurs du président américain, Joe Biden et Barack Obama, atteignent par ricochet tous les alliés de l’Amérique qui font front commun pour défendre un système de valeurs universel. les dirigeants des pays alliés de l’Amérique ont réagi comme un seul homme pour apporter leur soutien au président Zelensky, tandis que M. Orban et d’autres partisans de M. Poutine célébraient les propos par lesquels M. Trump faisait passer l’agressé pour l’agresseur. Renvoyé comme un serviteur, le président Zelensky est sorti de l’épreuve avec dignité. Avait il d’autres choix ? Que lui était il reproché ? D’avoir fait face sans ciller. D’avoir défendu les intérêts du peuple ukrainien, bien sûr. Il porte la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre leur patrie et celle des victimes de la destruction aveugle menée par le régime russe, mais pas seulement. Depuis trois ans, l’Ukraine défend les valeurs portées tant par l’Europe que par tous les pays qui se revendiquent de nos valeurs, à commencer par les États Unis d’Amérique. C’est une immense honte que Trump ait effectivement changé de camp dans la guerre russo ukrainienne en rejoignant la Russie. Les États Unis se sont alignés, non pas avec nos alliés de l’Otan, mais avec la principale menace historique de l’Otan : Moscou. Il est impensable qu’un président américain puisse agir ainsi. » Ce n’est pas moi qui le dis ; c’est John Bolton, qui fut nommé conseiller à la sécurité nationale au début du premier mandat de Donald Trump, après avoir été notamment sous secrétaire d’État sous George W. Bush.

tout comme M. Poutine pensait qu’il allait prendre le contrôle de ce pays en trois jours. Trois ans plus tard, la Russie s’épuise et ne paraît pas en mesure de gagner cette guerre, même en faisant appel à des troupes venant de Corée du Nord. Dans le même temps, l’Otan a vu la Suède et la Finlande la rejoindre.

L’Ukraine défend nos valeurs. Nous ne saurions accepter qu’on lui torde le bras pour accepter un accord de cessez le feu qui ne serait qu’un répit pendant lequel M. Poutine pourrait préparer la prochaine offensive.

Cette nouvelle orientation impliquera nécessairement de revoir nos priorités budgétaires pour augmenter encore significativement notre budget de défense. Comme l’ont rappelé les présidents Perrin et Kanner, « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Le chef d’état major des armées ne dit pas autre chose quand il annonce qu’il faut « gagner la guerre avant la guerre ». Les athlètes ne gagnent pas aux jeux Olympiques sans s’être préparés pendant des années. Il nous appartient de mobiliser sans attendre la population française, qui doit être pleinement consciente des menaces auxquelles nous sommes tous confrontés. La responsabilité de la sécurité et de la protection d’un pays repose collectivement sur toutes les personnes qui y habitent. Le gouvernement de la Suède a édité un livret envoyé à tous les habitants du pays. Ce document est destiné à aider la population à mieux se préparer pour tout ce qui peut arriver, que ce soient des accidents graves, des intempéries extrêmes, des cyberattaques ou des conflits militaires. Il y est indiqué que, si la Suède est attaquée par un autre pays, elle ne se rendra jamais, et que toutes les informations ordonnant de cesser la résistance seraient fausses. Ce message n’est pas inutile

J’ai remis hier, à Londres, une copie de ce livret au ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint Martin. Je souhaite vous le remettre également, monsieur le Premier ministre, afin que vous puissiez évaluer par vous même s’il ne serait pas pertinent de s’inspirer dès à présent de ces bonnes pratiques. vous l’avez dit avec raison, monsieur le Premier ministre, c’est à nous, Européens, de garantir la sécurité et la défense des Européens. Nos forces armées continentales, additionnées à celles du Royaume Uni, comptent plus de 2,5 millions de soldats professionnels, soit 25 % de plus que les forces russes, avez vous indiqué hier à l’Assemblée nationale.

J’ai pu le mesurer dans le domaine de la cybersécurité, où les hostilités ont démarré depuis bien longtemps. L’an dernier, pour faire face à l’ampleur de la menace cyber, la Maison Blanche m’invitait à Washington avec une délégation de parlementaires et d’experts français pour prôner la cybersolidarité.

C’est rassurant, car notre point faible est la fragmentation de notre organisation. L’État russe est connu pour chercher à utiliser la désinformation afin de nous diviser et d’altérer simplement notre force de résistance. C’est sa façon de chercher à gagner la guerre contre les démocraties sans avoir à utiliser la force militaire. C’est désormais un défi pour tous ceux qui défendent la liberté, la démocratie et les droits humains à chaque élection.

Les faits lui ont donné raison par le passé. Je suis persuadé que sa pensée doit continuer à nous guider, mes chers collègues. Si l’Europe se dote d’une puissance militaire à la hauteur de sa puissance économique,

Honte de l’humiliation subie vendredi dernier par le président ukrainien, qui, à la tête d’une nation se battant sans relâche depuis trois ans contre l’agresseur russe pour sa liberté, s’est vu inlassablement répéter qu’il n’avait pas les cartes en main.

aussi, face aux déclarations du président Trump, prenant à son compte le narratif russe au mot près, aux dépens de l’Ukraine et des Européens. La décision américaine de geler l’aide militaire à l’Ukraine est en ce sens une véritable trahison envers un pays allié et ami. Elle doit nous interroger sur notre capacité à prendre le relais des Américains en fournissant une aide immédiate et supplémentaire. Par cette décision, le président Trump veut forcer le président ukrainien et tout un peuple à capituler devant l’agresseur russe.

Les temps ont bien changé. Nous avons eu par le passé la conférence de Yalta. Aujourd’hui, nous venons de vivre la séquence stupéfiante de la Maison Blanche. Le monde libre est désormais incarné par les Européens. Devant le risque d’un grand effacement, il est temps de cesser de déléguer notre sécurité, de cesser de nous dénigrer alors que nous sommes puissants, et, surtout, de cesser de monnayer notre souveraineté. Nous devons lutter de toutes nos forces face au retour à une triste époque au cours de laquelle les grands empires dessinaient les frontières par la force tout en soumettant les peuples. Cette volonté américaine de vassaliser l’Europe et l’Ukraine en souhaitant imposer aux Ukrainiens une paix non concertée pour une guerre qu’ils n’ont pas provoquée doit agir sur nous comme un électrochoc. Comme la France le défend depuis 2017, l’Europe doit assumer elle même sa propre sécurité. Nous devons, en Européens, nous réarmer urgemment et faire face aux défis. La visite du Président de la République aux États Unis et le sommet pour l’Ukraine qui s’est tenu dimanche dernier à Londres ont marqué une étape importante. La France, la Grande Bretagne et l’Allemagne ont entraîné leurs partenaires à leur suite et elles ont su montrer au président Trump que l’Europe est unie et fédérée derrière une ambition commune.

si les agresseurs sont soutenus et si les Ukrainiens sont écartés des négociations. La paix que nous appelons de nos vœux devra respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. Nous souhaitons faire obtenir des garanties de sécurité fortes permettant de faire respecter un futur accord de paix sans lequel la Russie, comme par le passé, attaquera de nouveau l’Ukraine, voire un pays membre Conformément au plan préparé par la France et le Royaume Uni, le déploiement d’une troupe européenne sur le sol ukrainien peut être envisagé, mais uniquement après un accord signé. Cette « coalition de volontaires » devra prendre toute sa part au maintien de la paix. Si les Américains ne veulent pas y participer, alors il nous faudra élaborer ministre. Oui, nous venons de basculer dans une autre dimension. Les volontés impérialistes du président Poutine sur notre continent n’auront de limites que celles que nous serons en mesure de lui imposer. Il faut un sursaut européen et une initiative nouvelle.

Les déclarations du Premier ministre britannique et du chancelier allemand montrent qu’il y a enfin une prise de conscience de la nécessité de bâtir une force européenne indépendante des États Unis. En la matière, la France n’a pas à rougir.

En tant que seule puissance nucléaire de l’Union dotée d’une armée reconnue, notre pays est force d’entraînement pour créer les conditions de la sécurité de toute l’Europe. sur le partage de la dissuasion nucléaire doit être évoqué, mais il appelle des efforts de clarification afin d’éviter toute interprétation malencontreuse. Il est question non pas de déléguer à l’Union la dissuasion française, mais d’associer les pays européens aux exercices des forces de dissuasion. La décision ultime n’appartient naturellement qu’au seul chef de l’État français. La question du financement européen de notre effort de défense se pose. Nous devons être en mesure d’emprunter conjointement, sur le modèle de ce que nous avons déjà fait pour la covid 19, afin d’assurer la pérennité de notre continent. Dans un premier temps,

Je salue à ce titre les propositions de la présidente de la Commission européenne en vue de la mobilisation de près de 800 milliards d’euros pour la défense européenne, grâce à un assouplissement des règles budgétaires en faveur des investissements et à la mise à disposition d’une enveloppe de 150 milliards d’euros de prêts européens pour les membres de l’Union. Nous ne pouvons pas faire supporter l’entièreté de cet effort de guerre par les contribuables. Je suis donc favorable à l’utilisation des avoirs russes gelés pour armer et reconstruire l’Ukraine, mais aussi pour protéger l’Europe. il est clair que, avec le retour de la guerre commerciale entre Occidentaux, la construction européenne que nous avons bâtie sur un marché unique et une intégration économique forte entre États membres doit évoluer en profondeur.

la certitude que le bonheur des peuples ne peut exister que si nous défendons ce que nous avons de plus cher : la science avec la conscience, la justice, la démocratie et la liberté. Face à des partis d’extrême droite, partisans de Vladimir Poutine et soutenus par Elon Musk, qui se coalisent pour former une internationale réactionnaire en Europe, il est de notre devoir de défendre notre héritage. L’Europe que

dans laquelle 500 millions d’Européens demandent à 300 millions d’Américains de les défendre face à 140 millions de Russes, doit cesser. Ce n’est pas tant la supériorité économique ou militaire qui nous manque que la conviction d’être une puissance mondiale. L’Europe doit désormais se projeter comme étant cette puissance unie. C’est ce qu’elle a exprimé le week end dernier à Londres, au nez et à la barbe des autocrates et de leurs admirateurs. Opérons cette révolution copernicienne que le chef de l’État appelle de ses vœux depuis 2017. La parole La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

l’Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l’Ukraine risque d’être abandonnée et la Russie renforcée. Washington est devenue la cour de Néron : un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l’épuration de la fonction publique. C’est un drame pour le monde libre, mais c’est d’abord un drame pour les États Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d’être son allié puisqu’il ne vous défendra pas, puisqu’il vous imposera plus de droits de douane qu’à ses ennemis et vous menacera de s’emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du est en train de montrer ce qu’est l’art du à plat ventre. Il pense qu’il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d’accélérer les préparatifs de l’invasion de Taïwan. Jamais dans l’Histoire un président des États Unis n’a capitulé devant l’ennemi. Jamais aucun d’entre eux n’a soutenu un agresseur contre un allié, jamais aucun n’a piétiné la constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l’en empêcher, limogé d’un coup l’état major militaire, affaibli tous les contre pouvoirs, ou pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n’est pas une dérive illibérale ; c’est un début de confiscation de la démocratie. Rappelons nous qu’il n’a fallu qu’un mois, trois semaines et deux jours pour mettre à bas la République de Weimar et sa constitution. J’ai confiance dans la solidité de la démocratie américaine le pays proteste déjà. Mais, en un mois, Trump a fait plus de mal à l’Amérique qu’il n’en a fait en quatre ans lors de sa précédente présidence. Nous étions en guerre contre un dictateur ; nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Il y a huit jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison Blanche, les États Unis votaient avec la Russie et la Corée du Nord à l’ONU contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. Deux jours plus tard, dans le Bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie au héros de guerre Zelensky, avant de le congédier comme un palefrenier en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre. Cette nuit, il a franchi un pas supplémentaire dans l’infamie en stoppant la livraison d’armes pourtant promise. Que faire devant une telle trahison ? La réponse est simple : faire face Et d’abord ne pas se tromper : la défaite de l’Ukraine serait la défaite de l’Europe. Les pays baltes, la Géorgie, la Moldavie figurent déjà sur la liste. Le but de Poutine est le retour à Yalta, où fut cédée la moitié du continent à Staline. Les pays du Sud attendent l’issue du conflit pour décider s’ils doivent continuer à respecter l’Europe ou s’ils sont désormais libres de la piétiner. Ce que veut Poutine, c’est la fin de l’ordre mis en place par les États Unis et leurs alliés il y a quatre

effet, la vision trumpienne coïncide avec celle de Poutine : elle défend un retour aux sphères d’influence, les grandes puissances dictant le sort des petits pays. À moi, le Groenland, le Panama et le Canada ; à toi, l’Ukraine, les pays baltes et l’Europe de l’Est ; à lui, Taïwan et la mer de Chine… On appelle cela, dans les soirées des oligarques du golf de Mar a Lago, le « réalisme diplomatique »… Nous sommes donc seuls. Mais le discours selon lequel on ne peut résister à Poutine est faux. qu’affirme la propagande du Kremlin, la Russie va mal. En trois ans, la soi disant deuxième armée du monde n’a réussi à grappiller que des miettes d’un pays trois fois moins peuplé. Les taux d’intérêt à 25 %, l’effondrement des réserves de devises et d’or, l’écroulement démographique montrent que ce pays est au bord du gouffre. Le coup de pouce américain à Poutine est la plus grande erreur stratégique jamais commise lors d’une guerre. Le choc est violent, Le choc est violent, mais il a une vertu : les Européens sortent du déni. Exactement ! Ils ont compris en un jour, à Munich, que la survie de l’Ukraine et l’avenir de l’Europe sont entre leurs mains, et que trois impératifs

Cela coûtera cher. Il faudra donc en finir avec le tabou de l’utilisation des avoirs russes gelés. Il faudra aussi contourner les complices de Moscou à l’intérieur même de l’Europe, en formant une coalition des seuls pays volontaires, avec bien sûr le Royaume Uni.

Cette garantie passe par une force militaire suffisante pour empêcher toute nouvelle invasion. Enfin, et c’est le plus urgent, parce que c’est ce qui prendra le plus de temps, il faudra rebâtir la défense européenne, négligée au profit du parapluie américain depuis 1945 et sabordée depuis la chute du mur de Berlin.

C’est reconnaître que la France avait raison depuis des décennies en plaidant pour une autonomie stratégique. Il reste à la construire. Il faudra investir massivement renforcer le Fonds européen de défense, hors critères de Maastricht, harmoniser les systèmes d’armes et de munitions, accélérer l’entrée dans l’Union de l’Ukraine, laquelle possède aujourd’hui la première armée européenne, repenser la place et les conditions de la dissuasion nucléaire à partir des capacités française et britannique, et relancer les projets de bouclier antimissile et de satellite européens. Le plan annoncé hier par Ursula von der Leyen est un très bon point de départ. Et il faudra beaucoup plus. L’Europe ne redeviendra une puissance militaire qu’en redevenant une puissance industrielle. En un mot, il faudra appliquer le rapport Draghi, et pour de bon. Mais le vrai réarmement de l’Europe, c’est son réarmement moral. Nous devons convaincre l’opinion face à la lassitude et à la peur de la guerre, et, surtout, face aux comparses de Poutine, l’extrême droite et l’extrême gauche. Ces derniers ont encore plaidé hier, à l’Assemblée nationale, devant vous, monsieur le Premier ministre, contre l’unité européenne et la défense européenne. Ils disent vouloir la paix. Ce que ni eux ni Trump ne disent, c’est que leur paix, c’est la capitulation, la paix de la défaite, le remplacement de « de Gaulle Zelensky » par un « Pétain ukrainien » à la botte de Poutine, la paix des collabos qui ont refusé depuis trois ans toute aide aux Ukrainiens ? De la mésalliance atlantique ! Le risque est grand, mais l’humiliation publique de Zelensky et toutes les décisions folles prises depuis un mois ont fini par faire réagir les Américains. Les sondages sont en chute libre, les élus républicains sont accueillis par des foules hostiles dans leurs circonscriptions. Même Fox News devient critique ! Les trumpistes ne sont plus en majesté. Ils contrôlent certes l’exécutif, le Parlement, la Cour suprême et les réseaux sociaux, mais, dans l’histoire américaine, les partisans de la liberté l’ont toujours emporté. Ils commencent à relever la tête… Le sort de l’Ukraine se joue dans les tranchées, mais il dépend aussi de ceux qui, aux États Unis, veulent défendre la démocratie et, ici, de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l’Europe la puissance qu’elle fut un jour et qu’elle hésite à redevenir. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIsiècle. Vive l’Ukraine libre, vive l’Europe démocratique

monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 24 février 2025 a marqué le troisième anniversaire de la guerre d’agression menée par la Russie de Poutine contre l’État ukrainien. Je tiens ici à le rappeler avec force, cette agression militaire est injustifiable et constitue un crime, un crime contre le droit international et contre la paix. Dès lors, je tiens, au nom de mon groupe, à saluer et à exprimer ma profonde solidarité envers le peuple ukrainien, qui n’en peut plus de cette guerre. Depuis l’arrivée de Donald Trump, chacun pressentait que la donne allait changer, que les États Unis allaient mettre un terme à leur engagement.

pétrifié nombre d’États européens, qui n’avaient pas anticipé un tel retournement de situation. Nous fustigeons de telles méthodes qui violent les règles élémentaires de la diplomatie.

avons exigé le cessez le feu pour que l’intelligence triomphe de la bêtise de la guerre. Mais, lors de chaque débat, ici même au Sénat, c’est l’escalade militaire qui a emporté l’adhésion de la plupart des groupes, certains s’exprimant des accents guerriers qui, aujourd’hui, paraissent bien irresponsables au regard des centaines de milliers de morts et de blessés, ukrainiens ou russes. Tout cela pour en arriver où ? À la situation de 2014, mais avec un pays dévasté ! Je le dis clairement : ceux qui, depuis trois jours, font de la surenchère, appellent au surarmement et au développement de l’arme nucléaire,

à la domination américaine. Nous nous opposons frontalement à la démarche de Mme von der Leyen, laquelle veut consacrer 800 milliards d’euros au réarmement de l’Europe. Que cherchent ces gens ? La confrontation généralisée ? Quelle légitimité ont cette dame et la Commission européenne pour s’exprimer et agir de la sorte ?

La brutalité de Trump est une caricature de la puissance américaine et de la défense systématique de ses propres intérêts aux dépens de l’équilibre mondial. Rappelez vous le Vietnam, l’Irak, la Libye, et, plus récemment, la volte face en Afghanistan, sans oublier l’accompagnement, sans état d’âme, de la violence de Benyamin Netanyahou.

Cela montre bien que la voie du développement humain et de la concorde est, à l’inverse, dans le redressement des institutions internationales. Oui, mes chers collègues, nous sommes à un tournant, à un moment de rupture.

tant tardé, à œuvrer pour la paix, et non celui d’avoir plus fait la guerre ou livré davantage d’armes. Au printemps 2022, à Istanbul, Kiev a accepté de renoncer à adhérer à l’Otan et a confirmé son intention de ne pas se doter de l’arme nucléaire

en affirmant, au nom de l’Occident, que les Ukrainiens devaient « combattre jusqu’à ce que la victoire soit acquise et jusqu’à ce que la Russie subisse une défaite stratégique ». Johnson reprenait ainsi à son compte la logique d’affrontement imposée par les États Unis sur le sol européen depuis 1990.

aussi d’une hérésie stratégique. Quel est l’objectif ? S’agit il réellement de dissuasion ou préparons nous la reconquête des territoires annexés par la force à la Russie ? Nous refusons clairement l’envoi de troupes au sol pour poursuivre la guerre. Des soldats de la paix, oui ! De la chair à canon, non

Poussons à l’ouverture rapide de négociations avec toutes les parties concernées et, en particulier, les Ukrainiens

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le premier jour de l’agression russe contre l’Ukraine, les objectifs de Moscou sont aussi clairs qu’impitoyables

Vendredi dernier, jusque dans le Bureau ovale, le président Zelensky a résisté avec courage à ses deux inquisiteurs qui parlaient et, alors que le sang de milliers de jeunes coule encore aux portes de l’Europe. d’une mise en scène choquante, d’une insulte à l’histoire démocratique américaine et aux valeurs qui ont forgé le monde libre. Aujourd’hui, l’arrivée de l’administration Trump au pouvoir nous sidère. Devrait elle nous surprendre ? Non, le nouveau président américain n’a jamais caché son intention d’étendre son sur le plan diplomatique. Avant lui, rappelons le, le président Obama avait engagé un « pivotement » vers l’Asie, tandis que Joe Biden nous mettait en garde contre notre propension à croire dans les éternels dividendes de la paix. Certes, la méthode était moins brutale sous d’autres ères, mais, au fond, le message était identique à l’égard des Européens : il est temps de prendre en charge votre propre sécurité. Nous l’avons entendu. Aujourd’hui, n’oublions pas que derrière l’oncle Sam se cache le fantôme du Kremlin. Donald Trump nous a mis le pistolet sur la tempe, mais la menace est d’abord venue de l’Est, de la Russie impérialiste. Avant l’Ukraine, il y a eu la Géorgie et la Crimée. Demain, devons nous craindre pour les pays baltes ? Nous sommes en tout cas à un tournant historique. la pensée de Raymond Aron, l’immédiateté de la diplomatie ne produit pas de certitudes à long terme. Aussi, nous devons garder au moins un cap intangible, celui de tout faire pour garantir notre autonomie stratégique.

initiatives. Cependant, le Gouvernement doit clarifier sa position sur certaines propositions devant la représentation nationale. Je pense notamment à la possibilité de mobiliser l’épargne pour financer nos programmes de défense,

Il est par ailleurs urgent de relancer la réflexion autour du Livre blanc de la défense. Mobiliser l’ensemble de nos leviers économiques, en parallèle des initiatives de nos partenaires, c’est donner à l’Europe les moyens de disposer d’une puissance militaire pleinement dissuasive et véritablement souveraine. Pour s’engager dans cette voie, il faut évidemment que l’Europe arrête de douter. Elle est une grande puissance démographique, économique et militaire. Doit on pour s’en convaincre rappeler que la France, comme notre allié britannique, dispose de l’arme nucléaire ? Mon groupe aurait souhaité proposer autre chose aux jeunes générations que le projet d’une économie de guerre et un débat sur le partage du parapluie nucléaire. C’est triste et tragique, mais les valeurs qui nous sont chères, la liberté et l’humanisme, nous imposent de réagir. Ne pas douter ne suffit pas. Il faut également rester unis. Comme le disait François Mitterrand, « la France est notre patrie, l’Europe est notre avenir ». L’Europe en tant que véritable projet politique peine toujours à se concrétiser, car le continent européen résulte d’un mélange d’héritages et de différentes communautés de destin.

En ces moments d’inquiétude pour nos concitoyens, les forces républicaines doivent rester soudées et vigilantes face à une extrême droite qui absorbe facilement le narratif russe et réfléchit à sacrifier l’Ukraine sur l’autel d’une paix illusoire.

Tout cela n’exclut pas de conserver le lien transatlantique, aussi difficile que cela puisse paraître aujourd’hui. N’oublions pas qu’hier ce sont des milliers de soldats américains qui ont débarqué sur nos plages normandes et provençales au nom de la liberté. Comment imaginer que puisse être anéanti le sacrifice de ces jeunes venus sauver un pays qu’ils ne connaissaient pas ? En attendant, l’élan de solidarité envers l’Ukraine, affiché avec détermination ces derniers jours, est un signe d’espoir pour ceux qui croient en une Europe forte et souveraine. La déclaration du futur chancelier allemand appelant à une action commune va dans ce sens. Dans ces conditions, le RDSE partage la volonté du Gouvernement de réaffirmer le soutien de la France à l’Ukraine. Mais soyons lucides, rien ne se fera sans les Américains, et le président Zelensky restera maître de sa décision. L’Histoire nous a montré que les cessez le feu ne valent que par ceux qui les garantissent. À court terme, il me semble que notre responsabilité est d’aider les Ukrainiens à négocier au mieux avec l’axe opportun et immoral Washington Moscou.

d’un déploiement de forces européennes pour assurer la stabilité d’un potentiel cessez le feu est une option à ne pas écarter. Toutes les questions doivent être posées sans détour. Nous le devons à nos voisins roumains, moldaves ou polonais, qui se sentent en danger, sous la pression du pouvoir russe. Nos partenaires attendent de nous un signal clair. Ils espèrent que nous serons fidèles à nos valeurs et principes fondateurs et que nous garderons à l’esprit les mots de Rosa Parks : « Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. » La parole La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Monsieur le président, Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, il est des moments dans l’Histoire qui sidèrent le monde, des moments où chacun se souvient où il était et ce qu’il faisait. Le vendredi 28 février 2025 est indubitablement un de ces moments où l’Histoire s’écrit au présent. Le 28 février dernier, chacun a pu constater l’effondrement, en germe depuis des années, de l’ordre international issu de la guerre froide, du multilatéralisme et du droit international. Le 28 février, chacun a pu juger du glissement de la plus vieille démocratie du monde vers l’autoritarisme et le fascisme. Certains refusaient de le voir : ils sont tombés de leur chaise ! D’autres, dont nous faisons partie, l’annonçaient : ils ont tout de même reçu de plein fouet la violence de cette scène, tel un coup de poing dans l’estomac. Le 28 février, chacun a pleuré les valeurs de la démocratie et de la liberté, abandonnées par l’un des pays qui les avaient érigées en principe d’existence. Permettez moi de vous faire remarquer que les fascistes au pouvoir appliquent des politiques fascistes. La leçon vaut pour notre pays : lorsque l’on banalise les partis et les idées fascistes, lorsqu’on brocarde le droit et qu’on piétine la fraternité, on prépare l’effondrement d’une autre démocratie historique. Les États Unis d’Amérique seront ils encore une démocratie en 2028 ? Quelle que soit la réponse, cela change désormais peu de choses pour l’Europe. Au mieux, Washington n’est plus notre allié ; au pire, l’Amérique nous sera hostile. Le vertige saisit en prononçant ces mots. Cela étant, si l’humiliation du héros Volodymyr Zelensky, orchestrée par les médiocres ventriloques de Poutine, peut servir d’électrochoc à l’Union européenne, nous n’aurons pas tout perdu. L’extraordinaire dignité du président ukrainien, comme son extraordinaire courage, ainsi que celui de son peuple depuis le premier jour de l’agression russe, doit être notre boussole collective,

Ne nous y trompons pas : ce qui est attaqué par la Russie et, désormais, par les États Unis, c’est le principe même de l’Union européenne, à savoir une coopération entre États reposant sur le droit, la démocratie et la liberté. Ce qui est attaqué, c’est le potentiel politique et économique de l’Union. Pour résister à la vague des impérialismes américain, chinois et russe, nous n’avons d’autre choix que d’opérer un indispensable saut fédéral. Unie, l’Europe est en mesure de peser dans le nouveau désordre mondial et peut tenter de préserver ce qui peut encore l’être du droit international. Désunie, elle est condamnée à l’impuissance, voire à la dislocation, si aucune digue ne vient s’opposer

aucune paix ne sera possible dans un monde régi par les rapports de force entre empires. Il nous faut consentir à ces rapports de force pour préserver notre sécurité, nos valeurs et nos idéaux. Nous avons construit l’Europe pour éviter la guerre, mais il nous faut désormais préparer l’Europe face à la guerre. La position française, qui consiste à renforcer l’autonomie stratégique du continent, et la position historique des écologistes de bâtir une Europe de la défense trouvent aujourd’hui un nouvel écho. Nous appelons néanmoins l’exécutif français à se garder de tout triomphalisme et à remiser notre penchant national pour la vanité, cette même vanité qui nous a conduits à croire que nous pourrions raisonner Poutine et Trump. La période commande la modestie. Nous souscrivons à la nécessité de renforcer nos arsenaux, à l’idée d’exclure les dépenses militaires des critères de Maastricht, comme à la volonté d’un emprunt commun. Mais nous insistons sur la nécessité de communautariser davantage nos dépenses militaires, notamment nos achats, pour réaliser des économies d’échelle. En ce sens, la première mouture présentée par la Commission européenne, qui prévoit que plus de 80 % des efforts seraient réalisés par les États, ne nous satisfait pas.

Sacrifier nos services publics sur l’autel de notre défense conduirait la France au même destin électoral que les États Unis. Développer notre arsenal militaire pour le laisser entre les mains de dirigeants fascistes est un écueil que nous devons impérativement éviter. Ce qui vaut pour la France vaut naturellement pour toute l’Union européenne : celle ci doit préserver et amplifier ses politiques sociales. Nous entendons l’appel à élargir le parapluie nucléaire français au reste du continent

nous alertons sur la nécessité de conserver le cadre du traité de non prolifération et de ne pas nous livrer à une course aux ogives qui serait aussi dispendieuse que dangereuse. Les futures négociations de paix avec la Russie devront réenclencher le processus de désescalade des arsenaux nucléaires. L’autonomie stratégique européenne n’est pas qu’une question militaire. Elle ne peut être atteinte qu’en diminuant drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles et aux engrais azotés russes,

ce propos, monsieur le Premier ministre, est ce bien le moment d’encourir un incident diplomatique avec l’Algérie alors que nous cherchons à nous passer du gaz russe, qui fait couler le sang ukrainien, et du gaz azéri, qui fait couler le sang arménien ? L’économie de guerre est indissociable d’une écologie de paix. Il est donc impératif de préserver le Pacte vert et de sortir les investissements écologiques des critères de Maastricht. il nous faut poursuivre nos efforts pour mettre à bas les vecteurs de désinformation, de propagande fasciste et d’influence russe, au premier rang desquels le réseau social X. Le défi de l’autonomie européenne est colossal, mais nous avons les moyens de nos ambitions. Pour l’heure, notre urgence est la défense de l’Ukraine. À son peuple combattant, à son peuple sous les bombes, à son peuple en exil, nous réitérons l’expression de notre plein soutien et de notre entière admiration : les Ukrainiens

En tout état de cause, nous exigeons qu’aucun accord de cessez le feu – et,, de paix – ne soit conclu sans l’accord des représentants du peuple ukrainien et la participation de l’Union européenne. ! Un accord de cessez le feu devra inclure la libération de tous les prisonniers de guerre et civils ukrainiens détenus dans les prisons russes et exiger le retour des enfants ukrainiens déportés. Si l’Europe s’érige pour résister aux impérialismes, c’est pour faire prévaloir le droit et la paix, et pour être un point de repère et un appui pour l’ensemble du monde libre. La tâche est considérable, mais nous n’avons pas d’autre choix que de nous montrer

Cette guerre est pour l’Europe un retour à une dure réalité. Pendant soixante dix ans, l’Europe et la France se sont complu dans un rêve légitime : le droit international et la protection américaine garantiraient pour toujours la paix sur le continent. L’agression russe contre l’Ukraine a brutalement déchiré ce voile de certitudes. Trois ans plus tard, des négociations de paix semblent se dessiner, apportant leur lot non pas de soulagements, mais bien de nouvelles inquiétudes. L’est de l’Europe, trop de fois martyr, aiguise de nouveau l’appétit de la puissance impérialiste russe. Seule – ou presque –, la Pologne, chère à mon cœur, fortifie sa frontière orientale et craint légitimement l’avenir.

Une telle résolution du conflit apparaît particulièrement inquiétante pour la paix et la sécurité en Europe dans les années à venir. Elle entérine le droit du plus fort, la violation du droit international et le retour d’une diplomatie fondée sur la force brute et la domination des plus violents. Trois ans plus tard, nous devons également faire le bilan de l’action du Président de la République. Lorsqu’il va à Moscou en 2022 pour se concilier Poutine – où il se fait imposer une scénographie humiliante –, le Président de la République croit éviter la guerre. Résultat : les troupes russes attaquent l’Ukraine quelques jours plus tard. Il se rend alors à Kiev, où il assure Zelensky du soutien de la France et de son arsenal. Résultat : le verbe « macroner » est ajouté au dictionnaire ukrainien quelques semaines plus tard, avec comme définition : « parler beaucoup, n’agir jamais ». récemment, il se déplace à Washington où il s’affirme comme le chef de l’Europe face à un président américain imprévisible, tout en affichant sa bonne entente avec celui ci devant les caméras. Le soir même, Trump déclenche une guerre commerciale avec l’Union européenne. La diplomatie à la Macron est un fiasco qui se résume à flatter l’ego du Président de la République au prix d’humiliations à l’encontre de la France.

que ce qui se joue en Ukraine emporte des conséquences très lourdes pour la vie de notre pays et de nos territoires.

appelez les Européens à sortir du déni. Ils sont de plus en plus nombreux à le faire, y compris ceux qui étaient traditionnellement les plus atlantistes. En outre, vous pointez les fragilités des accords de Minsk

qui s’est rendu coupable de crimes de guerre en déportant des enfants ukrainiens,… Eh oui ! … ce qui lui vaut un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale. Vous évoquez

Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.

Une fois de plus, nous nous retrouvons dans cet hémicycle pour parler d’immigration : à croire que le sujet est quelque peu obsessionnel sur une partie de ces travées…

L’accord franco algérien de 1968 fixe les conditions de circulation, d’emploi et de séjour en France des ressortissants algériens. Ces derniers ne relèvent historiquement pas du droit commun, mais d’un régime dérogatoire, en raison des liens culturels et politiques noués de longue date Par plusieurs avenants, dont deux adoptés sous des gouvernements de gauche, le statut spécial des Algériens s’est progressivement rapproché du droit commun. Il reste plus favorable que celui ci sur certains points – je pense notamment au regroupement familial. Mais sur d’autres volets, comme les titres de séjour étudiants, Il est clair que l’attitude actuelle de l’Algérie vis à vis de la France n’est pas acceptable. Lorsque la France expulse légalement des ressortissants algériens condamnés sur son territoire, l’Algérie n’a pas à les refouler.

La France doit être ferme avec l’Algérie lorsqu’elle ne respecte pas nos accords. Le Président de la République et le ministre des affaires étrangères doivent dès lors engager un dialogue exigeant. les élus du groupe socialiste considèrent que la population algérienne n’a pas à payer pour l’attitude de son gouvernement. Aussi, nous sommes fermement opposés à la dénonciation unilatérale de cet accord. C’est d’ailleurs la position du Président de la République lui même, lequel a contredit son Premier ministre et son ministre de l’intérieur. Cette cacophonie au sommet de l’État est irresponsable. Même lors des véritables cohabitations, l’intérêt supérieur de la France a toujours conduit les deux chefs de l’exécutif à parler d’une seule voix sur les questions internationales. Le mauvais spectacle auquel nous assistons affaiblit la voix de la France sur la scène internationale, à un moment où notre pays doit y peser de tout son poids – le débat sur l’Ukraine vient de le montrer. Nos relations avec l’Algérie sont actuellement tendues – c’est une évidence – et les tensions vont bien au delà de la question migratoire. Voilà maintenant deux décennies qu’elles s’accumulent. La reconnaissance soudaine de la marocanité du Sahara occidental, sans aucun geste envers Alger, était une grave erreur de la part de la France.

de sa dénonciation unilatérale, c’est faire exactement ce que vous reprochez, à juste titre, au gouvernement algérien. Vous utilisez la rente mémorielle de notre douloureuse histoire commune à des fins de politique intérieure. tout ! Alors qu’il est indispensable de reprendre le dialogue, vous proposez, paradoxalement, de rompre un accord qui nous lie à l’Algérie depuis des décennies.

Cet accord est indissociable de l’histoire singulière qui lie la France à l’Algérie ; une histoire complexe, dont nombre de nos concitoyens sont les héritiers ; une histoire marquée par cent trente deux ans de colonisation, dont huit ans de guerre d’indépendance et six décennies de relations bilatérales sinueuses.

sans doute d’un relent colonial… À vos yeux, l’Algérie et les Algériens ne peuvent rien faire sans la France. Or, en cas de rupture, c’est la France qui a beaucoup à perdre. L’Algérie est un partenaire économique crucial pour la France, les échanges commerciaux entre nos deux pays atteignant 11,8 milliards d’euros en 2023. Que comptez vous dire aux 450 entreprises françaises installées en Algérie ? Aux 6 000 entreprises françaises qui y exportent des produits français ? Aux médecins algériens qui tiennent à bout de bras notre système hospitalier ? La dégradation de nos relations bilatérales a déjà provoqué une chute très importante des exportations françaises de blé vers l’Algérie, et le mouvement risque de s’accentuer. Que comptez vous dire à nos agriculteurs ? N’oublions pas non plus notre coopération sécuritaire avec l’Algérie, qui joue un rôle majeur contre le terrorisme dans la région du Sahel. Une fois encore, la pente dangereuse que vous suivez en courant après l’extrême droite nous conduit dans un mur. Vous prétendez protéger la France par des coups de force : en réalité, vous l’affaiblissez. Une histoire profonde lie nos deux pays. Permettez moi de reprendre les mots de Yazid Sabeg et Jean Pierre Mignard : « Des milliers de familles, des millions de personnes, quatre millions peut être de binationaux, d’enfants et de petits enfants, de parents algériens, ou à la fois algériens et français, vivent aujourd’hui dans un enchevêtrement d’appartenances, de souvenirs, de cultures, et forment une exceptionnelle mixité humaine. Ils sont la marque indélébile d’un destin partagé. Cette jeunesse issue de l’immigration algérienne, ancrée dans la République, désireuse à la fois de concilier son appartenance à la nation française sans répudier son algérianité, est le socle de notre avenir commun. Nos querelles la troublent et c’est injustifiable. Nous avons bien compris que c’est une réalité française que vous ne voulez pas voir. Dénoncer unilatéralement l’accord de 1968 ne la fera pas disparaître, bien au contraire ! Pour toutes ces raisons,

ce faisant, de construire un nouveau cadre de relations diplomatiques apaisées entre la France et l’Algérie, reconnaissant la complexité de notre histoire commune pour mieux la dépasser.

Ne laissez pas le ministre de l’intérieur faire des Algériens et de la relation franco algérienne les victimes de ses obsessions migratoires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1830, la France se lançait dans la conquête de la régence d’Alger qui était, depuis trois siècles, un territoire de l’Empire ottoman. deux années pendant lesquelles l’Algérie a été un territoire français et la guerre qui y a mis fin constituent l’histoire douloureuse que nos deux pays ont en partage. Six ans après la fin de la guerre de décolonisation, Paris et Alger ont conclu des accords visant à faciliter l’émigration des Algériens vers la France. Il est souvent dit que la France a fait cela pour satisfaire ses besoins en main d’œuvre. C’est juste, la France a offert aux Algériens des facilités pour venir dans notre pays, mais, il faut le rappeler, elle n’a forcé personne. Le fait que de nombreux Algériens aient choisi d’en bénéficier montre que ces accords ne leur sont pas défavorables. Il s’agit

Hélas, le gouvernement algérien continue de les altérer en ressassant inlassablement le passé colonial. En 2023, il a même réintroduit dans son hymne national un couplet demandant à la France de rendre des comptes.

C’est le gouvernement algérien qui est responsable devant son peuple ; la colonisation a eu son lot d’effets néfastes, mais ne peut pas tout expliquer. Le Vietnam a, lui aussi, été colonisé par la France lui aussi a obtenu son indépendance de haute lutte, après avoir affronté non seulement les Français, mais aussi les Américains, au cours d’un conflit majeur. Or, au cours des vingt dernières années, le taux de croissance du PIB algérien a été, malgré l’énorme rente gazière, bien inférieur à celui du Vietnam. La rente mémorielle, s’il fallait encore le démontrer, n’a jamais développé l’économie d’aucun pays. Tant que le gouvernement algérien instrumentalisera le passé pour dissimuler ou justifier ses propres lacunes, nos relations s’en trouveront dégradées. La dégradation fâcheuse de nos relations avec le gouvernement algérien a été récemment exacerbée par plusieurs événements. La France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Boualem Sansal est accusé d’avoir porté atteinte à l’unité nationale algérienne ; il est en réalité puni pour avoir tenu des propos déplaisant au gouvernement Une telle forme de censure n’honore pas du tout ce dernier et la France ne peut pas accepter que l’un de ses ressortissants soit ainsi détenu arbitrairement.

Parmi eux se trouvent quelques influenceurs douteux, dont certains appellent au meurtre, et une personne qui a commis un attentat terroriste à Mulhouse. Ces refus illégaux, puisque contraires au droit international, ont une conséquence logique, évidente la France doit s’interroger sur la suite des accords qui la lient à l’Algérie en matière d’immigration. Voilà deux ans déjà, Édouard Philippe attirait notre attention sur la nécessité d’un tel réexamen ; depuis lors, il a été rejoint par de nombreux responsables politiques. L’une des premières conditions de l’application du droit international est la réciprocité. Les refus du gouvernement algérien de permettre le retour sur son sol de ses ressortissants ne peuvent perdurer. Révisés plusieurs fois, ces traités peuvent être renégociés si cela est nécessaire. Nous considérons qu’ils doivent l’être, afin de mieux répondre aux impératifs auxquels sont confrontés nos deux pays. Nous souhaitons qu’un accord soit trouvé et que la relation entre nos deux peuples soit préservée, au mieux des intérêts de chacun.

de portée moindre, mais qui n’est pas anecdotique, celui du 10 juillet 2007, révisé le 16 décembre 2013. Ce traité prévoit une exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. L’accord facilite notre action diplomatique, mais il est devenu clair qu’il est plus avantageux pour les responsables algériens, compte tenu des liens personnels marqués que nombre d’entre eux ont en France ; ils l’utilisent pour faire des allers retours. Cet accord peut naturellement être mis sur la table dès lors que la coopération migratoire n’est pas satisfaisante.

monsieur le ministre, mes chers collègues, le 27 décembre 1968, la France et l’Algérie ont signé un accord définissant les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France.

de droit ; elle procède de la force brutale d’un régime autoritaire qui ne dit pas son nom, d’un régime qui affiche son antisémitisme en demandant à Boualem Sansal de récuser son avocat au motif que celui ci est juif, qui revendique son mépris envers les juifs, les harkis, les chrétiens et, plus largement, les Européens, notamment les Français. que dire des traitements discriminants et cruels qu’il inflige aux femmes, aux Berbères, aux Kabyles, sans oublier les campagnes racistes perpétrées par les médias d’État contre les migrants, notamment africains fait ! Dans ces conditions, pourquoi le Président de la République contredit il le Premier ministre et le ministre de l’intérieur, offrant ainsi au président Tebboune l’occasion de se jouer de nos divisions, y compris à la une de certains journaux algériens ? Pourquoi exprimer cette repentance perpétuelle, alors que nous ne récoltons en retour que mensonges historiques et humiliations, comme le Président de la République l’a appris à ses dépens et surtout aux dépens de la France, lorsqu’il a parlé de crime contre l’humanité ? Eh oui… Lorsque nous nous engageons sur ce chemin avec l’Algérie, il n’y a ni limite ni fin.

nous réclamons que le chef de l’État dénonce cet accord, non pas pour rompre définitivement toute diplomatie, mais pour reconstruire une relation sur de nouvelles bases – de fermeté, de respect et de réciprocité,

efficace et respectueuse. Mes chers collègues, il faut bien sûr lutter contre ceux qui portent la haine de la France, mais il ne faut pas oublier la main qui nourrit cette haine. Comme l’a justement indiqué Jean Sévillia, on « pourra regarder en face l’histoire de la présence française en Algérie […] le jour où l’opprobre ne sera plus jeté […] sur les Européens d’Algérie et les harkis et leurs descendants », le jour où une volonté de paix et de respect sera partagée sur les deux rives de la Méditerranée.

Compte tenu de ces difficultés, le Premier ministre a décidé, à l’issue de la réunion du comité interministériel de contrôle de l’immigration du 26 février dernier, qu’une liste d’individus serait soumise aux autorités algériennes, afin que ceux ci soient renvoyés d’urgence en Algérie, et que, à défaut d’une réponse favorable, nous réexaminerions l’ensemble des accords migratoires que nous avons avec ce pays. Il s’agit simplement de faire appliquer le droit et de défendre nos intérêts sur le plan migratoire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France et l’Algérie partagent un passé douloureux, qui, plus de soixante ans après l’indépendance algérienne, continue de susciter des tensions et des incompréhensions. La colonisation française en Algérie reste un sujet de crispation entre Paris et Alger. L’accord signé par les deux pays le 27 décembre 1968 réglemente la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens en France. Conçu à l’origine pour faciliter l’installation de travailleurs algériens sur notre territoire, il confère aux Algériens un régime dérogatoire au droit commun. Ces derniers bénéficient notamment de facilités d’entrée et de délivrance de titres de séjour, avec des durées allant jusqu’à dix ans. Cet accord, ciment des relations franco algériennes, suscite aujourd’hui de sérieuses interrogations. En 1968, il répondait à un besoin économique précis et annonçait un nouveau départ commun pour la France et l’Algérie. Depuis lors, le contexte a évolué et certains événements ont engendré une véritable crise diplomatique. En juillet 2024, l’Algérie s’est offensée du soutien exprimé par la France au plan d’autonomie marocain au Sahara occidental, territoire qui est le théâtre d’un conflit entre le Maroc et des indépendantistes soutenus par l’Algérie. En novembre dernier, l’écrivain Boualem Sansal, critique du régime algérien, a été arrêté à Alger. Qualifié par le président Abdelmadjid d’imposteur envoyé par la France, ce Franco Algérien à la santé fragile est toujours incarcéré, malgré les nombreuses demandes émanant de plusieurs pays. Enfin, le 3 février dernier, le président Tebboune a dénoncé le climat délétère entre l’Algérie et la France. L’attitude véritablement hostile des autorités algériennes vis à vis de notre pays est inquiétante. Dans ce contexte, il est tout à fait légitime d’évoquer les accords de 1968. Les facilités que la France accorde depuis des décennies aux Algériens semblent être en décalage avec l’attitude de l’Algérie, dont la coopération en matière d’immigration irrégulière est très insuffisante. Je souhaite évoquer ici le cas de l’assaillant qui a tué une personne et en a blessé d’autres le 22 février dernier à Mulhouse. Cet Algérien, arrivé illégalement sur le territoire français en 2014 et faisant l’objet d’une OQTF, est resté sur le sol français que l’Algérie a refusé à dix reprises de reprendre son ressortissant. Ce terroriste radicalisé et condamné plusieurs fois ne serait pas passé à l’acte sur le sol français si l’Algérie avait respecté son obligation de l’accueillir à la suite de son expulsion. Cet exemple fait écho à une autre situation qui a fait grand bruit en janvier dernier. Il s’agit bien entendu du cas de l’influenceur algérien Doualemn, expulsé légalement par la France vers l’Algérie le 9 janvier et renvoyé d’Alger à Paris le jour même. Les autorités algériennes bafouent ouvertement leur engagement envers la France ! Nous ne pouvons pas l’accepter ; c’est pourquoi, le 26 février dernier, lors de la réunion du comité interministériel de contrôle de l’immigration, le Premier ministre, François Bayrou, a défini une ligne claire la France ne doit pas continuer de distribuer des visas et d’accorder des facilités d’accès à son territoire aux ressortissants de pays qui ne respectent pas leurs propres obligations en matière migratoire. C’est pour cela qu’il a demandé aux inspections générales de la police nationale et des affaires étrangères de mener un audit interministériel sur la politique de délivrance des visas. Cette décision témoigne de la résolution et de la fermeté dont nous devons faire preuve envers les pays qui, comme l’Algérie, refusent de reprendre les ressortissants légalement expulsés du territoire français. Pourtant, en août 2022, les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune voulaient ouvrir une nouvelle ère dans les relations franco algériennes. Ils entendaient insuffler une nouvelle dynamique partenariale entre nos deux pays, afin de faire face ensemble aux nouveaux défis globaux et aux tensions internationales. Nous ne devons pas renoncer à toute relation avec l’Algérie. Nos deux pays doivent reprendre progressivement le dialogue pour remédier à la situation actuelle. Nous devons bien entendu maintenir une position de franchise et de fermeté. L’Algérie doit respecter ses obligations envers la France, sans quoi nous serons dans notre droit de prendre de nouvelles mesures nous permettant de respecter notre souveraineté en matière migratoire. La conjoncture est d’autant plus dommageable qu’elle bafoue le passé que nous avons en commun. Celui ci est complexe, marqué par des blessures encore vives, mais aussi animé par des liens humains et culturels indéniables. Acteurs d’une histoire commune, nos deux pays ont tissé des rapports étroits, notamment sur le plan mémoriel, comme en témoigne le travail mené par la commission Stora à la fin de l’année 2024. Nos liens économiques ont également été renforcés depuis le début de la guerre en Ukraine. À titre d’exemple, les exportations algériennes d’hydrocarbures vers la France avaient augmenté de 15 % en 2023, en raison de la volonté française de réduire sa dépendance au gaz russe. Nous devons, par la reprise du dialogue diplomatique, trouver une nouvelle manière de collaborer avec l’Algérie, sans renier nos engagements ni nos principes. Veuillez conclure, ma chère collègue. Il nous appartient de définir un cadre juste, équilibré et respectueux de la souveraineté de chacun.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie sont avant tout le fruit de surenchères politiques et médiatiques qui cherchent à capter l’attention à des fins électorales. Je m’interroge alors : quel est le véritable objectif ici ? Faut il raviver une guerre d’Algérie au travers de tensions artificielles pour des raisons politiciennes ? Nous devons être extrêmement vigilants face à de telles dérives. À ce propos, permettez moi de citer une déclaration célèbre de l’évêque d’Oran : « La France et l’Algérie n’hésitent pas à se blesser mutuellement. L’originalité de ces blessures est qu’elles sont de celles que ne peuvent s’infliger que de véritables amis. » Le ministre des affaires étrangères a récemment déclaré : « Si un pays ne coopère pas avec les autorités françaises, je vais proposer que tous les pays européens en même temps puissent restreindre leurs délivrances de visas. » Une telle déclaration, déconnectée des réalités diplomatiques, mérite d’être mise en perspective. Elle témoigne d’une vision simpliste et unilatérale, qui oublie que les relations internationales se bâtissent sur le respect et la coopération, non sur la pression ou les menaces. L’accord franco algérien de 1968, dont il est notamment question ici, loin d’être un privilège, est le fruit d’une histoire partagée, marquée par des luttes, des sacrifices et des réconciliations. Il a permis à des milliers de familles de contribuer à la richesse de notre nation. Pourtant, force est de constater que cet accord, bien qu’il ait joué un rôle crucial dans le passé, n’est plus aujourd’hui qu’une coquille vide.

Le débat sur sa révision est donc, en réalité, un faux débat. L’Algérie est un acteur clé dans sa région et sur le continent africain. Elle possède des ressources propres et une politique indépendante. Il est dans l’intérêt de nos deux deux pays de maintenir une coopération pragmatique, en particulier dans des secteurs comme celui de la santé, des médecins algériens permettant de combler les pénuries dans les déserts médicaux. De plus, l’Algérie représente un marché important pour nos exportations et reste un partenaire stratégique en Afrique du Nord et au delà. C’est enfin la coopération en matière de sécurité et de renseignement entre nos deux nations que nous devons préserver. Alors, derrière cette escalade, nous le savons, il y a des stratégies électorales. Certains acteurs politiques, conscients de l’imminence des échéances électorales de 2027, cherchent à maximiser leur influence au sein de leur parti et à se poser en défenseurs de l’identité nationale. cette attitude, cette volonté de jouer avec les peurs, n’est pas à la hauteur de ce que nous attendons d’une politique étrangère responsable. Cette politique de confrontation n’a que trop duré. Nous devons arrêter ce jeu dangereux qui consiste à instrumentaliser la question de l’immigration pour des raisons purement électorales. À ce sujet, la position du Président de la République mérite d’être soulignée. Emmanuel Macron a, enfin, pris ses responsabilités, marquant la fin de la récréation diplomatique. Il a clairement sifflé la fin du jeu en soulignant notamment que l’« on ne peut pas se parler par voie de presse », et que les relations entre la France et l’Algérie ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques. Il a également rappelé que des millions de Français, nés de parents algériens, « vivent en paix, adhérant aux valeurs de la République Enfin, je tiens à citer les propos de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États Unis et ancien représentant permanent auprès des Nations unies ; il a indiqué avec clairvoyance : « Tôt ou tard, nous conclurons que la politique suivie vis à vis de l’Algérie nous mène dans une impasse. On fera appel aux diplomates pour réparer le gâchis. » Ces mots doivent résonner comme un avertissement. Il est grand temps de sortir de cette impasse et de reprendre un dialogue constructif, loin des polémiques inutiles. Il est impératif que nous mettions de côté nos ambitions électorales et agissions dans l’intérêt de notre pays, mais aussi de la stabilité et de la coopération internationales. Nous avons la responsabilité de rétablir une diplomatie respectueuse, fondée sur le respect de nos engagements mutuels. Je vous invite à reconsidérer toute approche punitive et à favoriser une diplomatie pragmatique et constructive. Nous avons la responsabilité de remettre l’intérêt national au cœur de nos décisions. La parole

le dialogue, la diplomatie. Il s’agit simplement d’avoir les instruments nécessaires pour défendre collectivement nos intérêts, en Européens. C’est aussi cette volonté d’avoir une Europe souveraine, maîtrisant ses frontières, qui est au cœur de la diplomatie française portée par le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat public s’est emparé du sujet des relations franco algériennes dans un contexte dramatique.

La détention arbitraire du franco algérien Boualem Sansal ou encore les affaires récentes concernant les soi disant influenceurs sont autant de signes actuels et convergents qui nous sont envoyés par le pouvoir algérien. Le Président de la République aura pourtant essayé de renouveler nos relations avec l’Algérie. Malgré tous ses efforts, sa démarche visant à les normaliser aura largement été vaine, Nous connaissons tous les vicissitudes des relations entre l’Algérie et la France. Nous savons également l’importance des liens humains entre nos deux pays : 650 000 Algériens vivent en France et 30 000 Français résident en Algérie.

Quant à l’accord de 2007, encore étendu en 2013, qui tend à dispenser de visa les détenteurs de passeport diplomatique ou de service, sa suspension me semble devoir être directement envisagée et aurait le mérite de ne concerner que les cadres du régime. Rien ne vient plus justifier une faveur de cette nature dans les circonstances actuelles. Rapprocher la situation algérienne du droit commun en matière migratoire et de droit au séjour serait tout simplement l’expression de notre volonté souveraine de réduire les flux d’entrée sur le territoire national.

nous le savons, l’importance globale de ces derniers ne nous permet plus d’accueillir ni d’intégrer les primo entrants conformément à notre modèle républicain. L’accord franco algérien de 1968 a mis en place entre nos pays un régime dérogatoire au droit commun dans le domaine migratoire.

Depuis 2022, nous attendons d’ailleurs la négociation d’un quatrième avenant. Il faut garder à l’esprit que l’immigration en provenance de ce pays se distingue des autres flux par son volume. Bien loin d’être une « coquille vide », comme l’a pourtant qualifié le président Tebboune, l’accord de 1968 a entraîné la délivrance par la France de plus de plus de 250 000 visas et de 30 000 nouveaux titres de séjour à des Algériens en 2024. Aujourd’hui, un titre primo délivré sur dix l’est à un ressortissant de ce pays, tandis que les certificats de résidence concernant les Algériens représentent 15 % du stock global des titres valides.

l’Algérie ne fournit pas le surcroît de coopération dans la lutte contre l’immigration illégale que nous pourrions légitimement attendre, mais elle ne respecte même pas ses obligations internationales. Bien avant la reconnaissance de la détérioration de nos relations bilatérales en 2024, l’Algérie manifestait déjà sa très mauvaise volonté lorsqu’il s’agissait

En 2024, moins de 10 % des Algériens expulsables ont pu être renvoyés dans leur pays, soit près de 3 000 personnes sur 33 754 interpellations pour infraction à la législation sur les étrangers. Je conclurai en évoquant l’organisation de notre diplomatie migratoire. Au cours de la mission sénatoriale qui vient de s’achever, 197 instruments internationaux ont été recensés dans le domaine migratoire. De nature, de portée et d’intérêt très variables, les accords applicables représentent une belle sédimentation, voire un joli « fouillis » – nous les avons qualifiés ainsi –, et ne forment aucunement une politique cohérente, dont nous avons pourtant besoin. Nous avons également identifié, avant même la polyphonie gouvernementale sur l’accord de 1968, une réelle différence d’approche entre le Quai d’Orsay et Beauvau. Elle dure depuis bien longtemps et dépasse donc les actuels titulaires de ces fonctions. Aujourd’hui, nous appelons de nos vœux une meilleure structuration de notre diplomatie migratoire, notamment un fonctionnement plus régulier du comité interministériel de contrôle de l’immigration, qui ne s’était pas réuni au niveau des ministres depuis 2023. La parole est à M. le ministre délégué.

lamentable ! Nous sommes confrontés, en réalité, à une stratégie délibérée visant, d’une part, à saturer l’espace médiatique autour des enjeux d’immigration

en France, ou à cette ancienne tête de liste aux élections européennes, qui déclarait avant hier que l’Algérie « a du sang sur les mains ». En somme, tout cela constitue une escalade dangereuse,

Fondée sur une avalanche de contrevérités, ensuite, parce qu’elle vise à faire croire que les accords de 1968 auraient ouvert les vannes de l’immigration algérienne, alors que ceux ci visaient précisément à la limiter.

aucune exécution d’OQTF supplémentaire. Quand on est ministre, on est jugé sur ses résultats. En l’occurrence, cette montée des tensions a t elle permis d’obtenir quoi que ce soit de la part du gouvernement algérien ? Absolument rien

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, inscrire ce débat à l’ordre du jour dans un contexte marqué par des manœuvres politiciennes opportunistes n’est ni sage ni responsable. Les polémiques de ces dernières semaines ont blessé de nombreux Français ayant un lien affectif avec l’Algérie. Ces femmes et ces hommes, véritables ponts entre nos deux pays, ont éprouvé une légitime indignation. Quant aux nombreux Algériens qui vivent et travaillent en France et contribuent à la richesse de notre pays, beaucoup se sont sentis stigmatisés, instrumentalisés et méprisés. Je pense notamment aux médecins algériens – c’est la première nationalité étrangère exerçant dans les hôpitaux français – qui font fonctionner un système de santé à bout de souffle. Obsession de l’extrême droite et désormais du Gouvernement, l’accord de 1968 cristallise toutes les tensions. Cet accord a pourtant été révisé à trois reprises : chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ces évolutions ont toujours eu lieu dans la discrétion, loin de toute agitation médiatique, et dans un esprit de respect mutuel. Aujourd’hui, largement vidé de sa substance, l’accord constitue un frein aux droits des Algériens, les excluant de toutes les avancées législatives et administratives dont ont bénéficié d’autres ressortissants étrangers. Par exemple, les Algériens ne peuvent pas prétendre aux cartes « compétences et talents », instaurées en 2006, qui facilitent l’installation des travailleurs hautement qualifiés, tels que les médecins et les ingénieurs. Autre inégalité frappante : les étudiants algériens, contrairement à d’autres nationalités, sont soumis à une obligation d’autorisation de travail, compliquant considérablement leur accès à l’emploi et freinant leur insertion professionnelle. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le discours ambiant autour de cet accord de 1968 relève plus du fantasme que de la réalité. Il y a, d’un côté, la propagande politique et, de l’autre, le droit, comme l’a d’ailleurs rappelé le tribunal administratif de Melun. nous devrions revenir une nouvelle fois sur cet accord, optons pour la retenue, le respect mutuel et la diplomatie ! En lieu et place, le Gouvernement a choisi l’escalade verbale, l’outrance et le tapage médiatique. Ainsi, nous voyons une frange de la classe politique française, soucieuse de ses ambitions personnelles, sacrifier l’axe Paris Alger sur l’autel de calculs électoralistes à courte vue. Cette surenchère a libéré une parole algérophobe qui se traduit par le mensonge, la menace et un négationnisme historique indigne de notre époque. Nous assistons depuis plusieurs semaines à une dérive inquiétante. Pensant à tort que la polémique fait une politique, voire une géopolitique, des ministres affirment que la colonisation de l’Algérie aurait eu des aspects positifs, tandis que le fils d’un ancien Président de la République appelle à incendier l’ambassade d’Algérie, sans que cela émeuve outre mesure le Gouvernement. De son côté, le Premier ministre multiplie les sommations et les ultimatums. Faisons nous face à une « trumpisation » de la classe politique française ? Assistons nous à la libération d’une algérophobie latente, nourrie par des clichés coloniaux et par un ressentiment anti algérien, toujours aussi vivace dans certains esprits ? ? S’agit il de donner des gages au Rassemblement national, dont dépend la survie de ce gouvernement ? Hélas, il semble bien que ces trois explications se conjuguent, révélant une dérive préoccupante dont les conséquences pourraient être durables pour les relations franco algériennes. J’ai toujours été engagé en faveur d’un rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Je suis convaincu que l’axe Paris Alger peut se construire sur l’exemple de l’axe Paris Berlin. cette relation doit être refondée sur la vérité, la justice et le respect mutuel. Pour ce faire, il faut cesser cette reconnaissance mémorielle au compte gouttes, dictée par les calculs politiciens du moment. En effet, l’histoire ne s’efface ni ne se maquille au gré des opportunités électorales. Elle doit être assumée dans sa globalité, avec courage et lucidité. Clemenceau lui même, pourtant homme de son temps, dénonçait déjà les massacres commis en Algérie en déclarant : « Nous avons rempli l’Algérie de ruines et de cendres, nous avons à répondre de milliers d’hommes massacrés. » Ce constat dressé il y a plus d’un siècle reste d’une actualité criante face aux tergiversations de notre pays sur son passé colonial. Il est temps que certains réalisent – enfin ! – que le seul bienfait de la colonisation fut la décolonisation. Ne vous en déplaise ! Mes chers collègues, nous nous approchons dangereusement du point de non retour. Hier, nous nous sommes brouillés avec le Mali, la faute revenant, nous a t on dit, au gouvernement malien.

Deux hypothèses s’imposent : soit nous sommes des génies incompris, détenant seuls la vérité face à un continent entier, soit nous avons un sérieux problème dans notre manière d’aborder nos relations avec les nations africaines souveraines. Pendant que nous accumulons les brouilles et les malentendus, d’autres pays avancent. d’autres pays avancent. Conscients des mutations du monde, ceux ci travaillent à bâtir des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel et le principe du partenariat gagnant gagnant. Je ne vous parlerai pas du plan Mattei de l’Italie… L’Algérie accueille près de 450 entreprises françaises sur son territoire tandis que plus de 6 000 autres profitent des exportations françaises vers ce marché. Dans ce battage politico médiatique, avons nous mesuré les répercussions potentielles sur ces entreprises et les milliers d’emplois qu’elles créent ? Dans le nouvel ordre international qui se dessine, il ne suffit plus, monsieur le ministre, d’imposer, de sermonner ou de mépriser. Il faut écouter, comprendre et construire des alliances solides. Concluez ! Si nous persistons à voir l’Afrique comme un théâtre où nous seuls dictons les règles du jeu, nous ne ferons que précipiter notre déclassement. Le monde change, les rapports de force évoluent et il serait temps d’adapter notre logiciel diplomatique avant qu’il ne soit trop tard. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me tiens devant vous en éprouvant un sentiment d’urgence républicaine. En effet, les événements récents entre la France et l’Algérie nous plongent dans une crise sans précédent. Celle ci va, à mon sens, bien au delà

car nous devons faire face à une série de dérives qui atteignent le cœur de notre cohésion nationale, notre sécurité et notre souveraineté, comme d’autres

Boualem Sansal, qui se meurt dans les geôles du régime d’Alger tout simplement parce qu’il est un peu trop libre ou qu’il aime trop la France : ces deux tragédies récentes illustrent, en réalité, un problème bien plus large et bien plus profond. Ces drames sont, en fait, les symptômes d’un échec massif de la gestion de nos flux migratoires. Cette crise trouve en l’Algérie l’un de ses aspects les plus visibles. En 2025, plus de 2,5 millions de personnes d’origine algérienne vivent en France, un nombre en constante augmentation.

ne font qu’accentuer une situation déjà critique, car, dans le même temps, 33 000 Algériens ont été contrôlés en situation irrégulière en France en 2023, dont seuls 3 000 ont fait l’objet d’une procédure d’éloignement. Ce décalage entre réalité des contrôles et mise en œuvre des expulsions illustre bien l’inefficacité de notre politique actuelle. Mon propos n’est pas de stigmatiser le peuple algérien, qui, comme nous tous, aspire à la paix et à la prospérité. La source du problème, à laquelle il faut s’attaquer, est le régime algérien, régime autoritaire qui a failli à ses responsabilités en laissant prospérer une immigration incontrôlée et en ne régulant pas les flux sortant de son pays. C’est à lui qu’il faut demander des comptes ! Pour cela, l’a indiqué le ministre de l’intérieur, il nous faut adopter une réponse graduée en commençant par des mesures individuelles. D’abord, il faut identifier les ressortissants algériens les plus dangereux pour les expulser vers leur pays d’origine dans les meilleurs délais. il ne faut pas s’interdire de s’interroger sur le bien fondé des accords de 1968 et de 2007. ne pouvons pas non plus faire l’économie d’une réflexion sur l’automaticité de la délivrance des visas. Chaque visa délivré devrait, à mon avis, correspondre à l’expulsion effective d’un ressortissant sous OQTF. la réflexion pourrait se porter sur la suspension des flux financiers des Algériens de France vers l’Algérie ou sur l’aide au développement. En tout état de cause, nous devons démontrer au régime algérien que la France ne peut plus ouvrir sa porte à ceux qui veulent abuser de notre générosité. La parole

Le « front diplomatique » que le ministre d’État, ministre de l’intérieur appelle de ses vœux est un oxymore, car la diplomatie consiste à négocier la paix par le dialogue. Le contre exemple américain nous le confirme. Pourtant, nous comprenons aisément les raisons de l’ire du ministre, que beaucoup partagent sur ces travées. L’actualité nous a encore montré le peu de cas que le régime algérien fait des accords qui nous lient. Il faut,

L’Algérie doit rester un partenaire économique ouvert aux exportations françaises, lesquelles représentent 4,5 milliards d’euros par an, un chiffre en nette baisse.

Chaque matin, Radya Rahal, présidente du conseil consulaire à Alger, m’envoie, comme à Olivier Cadic, les gros titres de la presse algérienne. Après s’être interrogés sur une désescalade ce week end, ces médias soulignent ce matin la cacophonie des gouvernants français. En Algérie, plus de 30 000 Français sont inscrits au consulat. Quelque 400 entreprises françaises sont installées là bas. Régulièrement, Mme Rahal m’indique les inquiétudes de la communauté française à Alger,

Merci

Les autorités algériennes continuent de considérer cet accord comme un droit acquis hérité de l’histoire. Or cette situation ne semble plus acceptable aujourd’hui. Une politique migratoire plus restrictive est réclamée par nos compatriotes et semble s’imposer. En 2024, la France a délivré 336 000 titres de séjour près de 160 000 demandes d’asile, soit près de 500 000 entrées sur notre territoire. Dans le contexte de tensions migratoires que nous connaissons, l’accord franco algérien, signé il y a plus de cinquante ans, apparaît désormais anachronique. En matière d’immigration, nous devons par ailleurs harmoniser le droit français avec le droit européen en tendant vers une plus grande cohérence. Or le régime dérogatoire actuel fait obstacle à cette volonté de régulation et de fermeté. Je citerai par exemple l’accès à un certificat de résidence de dix ans après seulement trois ans de séjour, contre cinq ans pour d’autres nationalités, ou encore les conditions d’admission au titre du regroupement familial, qui sont assouplies sans vérification stricte des conditions d’intégration. Enfin, la question la plus conflictuelle est le manque de coopération – c’est une litote ! – de l’Algérie dans la délivrance des laissez passer consulaires, compromettant le retour dans leur pays

Plus grave encore, un ressortissant algérien a tué un homme et blessé cinq personnes dernièrement à Mulhouse ; cet homme, présent illégalement en France depuis 2014, sortait de prison où il avait effectué une peine pour apologie du terrorisme. Nous avons appris, appris, depuis, que ce meurtrier avait été présenté dix fois sans succès aux autorités algériennes. Aussi, face à l’intransigeance des autorités algériennes en matière de laissez passer consulaires, la France doit elle instaurer instaurer un rapport de force. Cela peut passer par une remise en cause de l’accord de juillet 2007 qui vise à faciliter les déplacements officiels de courte durée pour les détenteurs de passeports diplomatiques ; cela peut aussi signifier restreindre, voire bloquer, la quantité de visas délivrés, comme l’a préconisé François Noël Buffet. Le rapport de force peut enfin passer par la dénonciation ou la renégociation de l’accord de 1968. Une telle dénonciation unilatérale semble justifiée juridiquement ; elle est en tout cas possible en s’appuyant sur la convention de Vienne sur le droit

a fait preuve d’une moindre clarté : il a affirmé qu’il ne dénoncerait pas de manière unilatérale les accords de 1968, arguant qu’un tel acte risquerait d’« envenimer inutilement les relations avec l’Algérie ». Il a préféré concentrer son attention sur l’avenant de 1994, suggérant que des ajustements étaient possibles. La dénonciation de cet

je sais les risques qu’il y a à faire attendre le sénateur Karoutchi, mais aussi à le laisser parler en dernier… Du fait d’une histoire partagée qui a créé des liens complexes, mais profonds entre nos deux pays, l’Algérie est le premier pays d’immigration en France. C’est aussi, après la Chine et le Maroc, le troisième pays auquel nous accordons le plus grand nombre de visas. Il est donc bien naturel, dans un moment où les pouvoirs publics, la demande de nos concitoyens, s’attachent à mieux contrôler les flux migratoires, d’évoquer sans tabou la question des accords franco algériens relatifs à la circulation des personnes. Et je voudrais remercier les sénateurs qui d’organiser aujourd’hui ce débat. Je crois toutefois important de distinguer deux problématiques, comme je l’ai fait tout à l’heure lors du débat. La première est celle des reconduites dans leur pays de ressortissants algériens ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. À cet égard, l’Algérie relève pour l’essentiel du droit commun, précisé par le protocole du 28 septembre 1994 portant accord de coopération en matière de délivrance des laissez passer consulaires, et non d’un accord dérogatoire. Nous rencontrons, pour procéder à des éloignements, des difficultés significatives, qui ne sont malheureusement pas propres En 2024, je le mentionnais, 41 % seulement des laissez passer consulaires demandés à Alger ont été délivrés dans les délais utiles. Ce chiffre, bien qu’en augmentation, reste bien sûr insuffisant. Les conséquences de ces difficultés peuvent être dramatiques, comme nous l’avons constaté avec l’attentat de Mulhouse, commis par un ressortissant algérien déjà condamné, radicalisé, et dont nous avions demandé l’éloignement à plusieurs reprises, en vain, aux autorités algériennes. Plus récemment, dans un contexte de tensions bilatérales renforcées, nous avons été confrontés à des difficultés spécifiques concernant des ressortissants algériens disposant de documents d’identité en règle,

de la clarté pour faire entendre nos intérêts, renégocier ces accords et faire respecter nos objectifs de politique migratoire. Voilà qui m’amène à la deuxième problématique, celle des accords bilatéraux en matière de circulation de personnes.

messieurs les sénateurs, que cet accord facilite l’immigration familiale au détriment de l’accueil de talents, d’étudiants ou de professionnels. Il est également moins exigeant que le droit commun en matière de vérification de l’intégration des immigrés. Il ne correspond donc ni aux exigences du temps présent

le champ de la lutte contre l’immigration irrégulière. La position du ministère est en conséquence de plaider pour une renégociation qui aurait, je le disais tout à l’heure, un triple objectif : rapprocher le régime s’appliquant aux Algériens du droit commun, notamment en matière d’immigration familiale introduire des dispositifs attractifs pour les profils les plus dynamiques ; renforcer les exigences républicaines d’intégration, qu’elles soient linguistiques ou civiques. Une telle renégociation n’aurait rien de nouveau, puisque l’accord a déjà été modifié à trois reprises, en 1985, en 1994 et en 2001. En 1994, par exemple, nous avons rendu obligatoire la présentation d’un passeport et d’un visa pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Vous le voyez, on a donc su faire évoluer de façon

J’ai mentionné aussi tout à l’heure – c’est un point important – l’accord du 10 juillet 2007, révisé en 2013, qui prévoit l’exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service. Nous avons pris, sur la base de cet accord, des mesures restrictives, en durcissant sa mise en

franco algérienne ; il est, bien sûr, de faire respecter nos intérêts, de faire entendre nos exigences et d’assumer le rapport de force avec les représentants de la nomenklatura. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai essayé de vous exposer

et une culture du résultat », avec pour seule boussole l’intérêt de la France et des Français. Nous n’aurons, et nous n’avons, aucune difficulté à assumer des rapports de force là où c’est utile et à utiliser la large palette d’instruments dont nous disposons

Chaque État est libre, et c’est heureux, de gérer ses affaires, de gérer la manière dont il envisage la politique migratoire.

Faites respecter la France, faites respecter les accords internationaux, et tout ira bien. Si l’Algérie respecte les accords, très bien ; si l’Algérie ne les respecte pas, la France, elle, se fera respecter.

Merci